Territoires. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Face à l'épisode de gel d'une ampleur sans précédent qui touche depuis une semaine une large partie de la France, je souhaiterais tout d'abord adresser toute ma solidarité aux paysannes et aux paysans qui ont perdu, en une nuit, les fruits d'une année de travail. Des vignobles du Chablis aux arboriculteurs de la Drôme, en passant par les semis de betteraves de la Seine-et-Marne, c'est la désolation. Cette catastrophe ne peut être prise comme un phénomène isolé. phénomène isolé. Elle est bien évidemment liée au dérèglement climatique. Elle fait suite à de nombreux précédents, et ce type d'aléa se reproduira à un rythme difficilement soutenable pour la pérennité du régime actuel d'indemnisation. Le déclenchement de la procédure de calamité agricole et son déplafonnement étaient bien sûr indispensables, mais ce système n'est plus adapté pour faire face à ces épisodes climatiques extrêmes à répétition il faut attendre de longs mois pour être indemnisé, ce qui ne permet pas de maintenir à flot des trésoreries déjà exsangues. Les critères d'éligibilité pour accéder à ce fonds sont drastiques, avec un seuil qui évince un grand nombre de petites exploitations, sans compter toutes celles qui en sont totalement exclues. Les viticulteurs doivent recourir à des assurances privées, inadaptées et coûteuses. Il faut maintenant engager des mesures structurantes à même de couvrir tous les risques climatiques pour toutes les cultures. L'excellent rapport sénatorial de Nicole Bonnefoy constitue une bonne base de réflexion Monsieur le ministre, votre prédécesseur Didier Guillaume s'était engagé, voilà plus de deux ans, à remettre à plat le régime de calamité agricole. Les travaux ont-ils avancé depuis lors

Comme je l'ai souligné voilà quelques jours, cet épisode exceptionnel a donné lieu à la plus grande catastrophe agronomique du début du XXI siècle. Songez, mesdames, messieurs les sénateurs, que des centaines de milliers d'hectares

monsieur le ministre. Cet épisode nous rappelle aussi combien notre modèle agricole hyperspécialisé, trop souvent en monoculture, est très fragile face au changement climatique. Les politiques publiques doivent soutenir et financer des modèles agricoles plus résilients ; c'est une priorité.

L'actualité l'a encore montré, les start-up ont réussi à terrasser les géants de l'industrie pharmaceutique en matière d'innovation contre la covid-19 : alors que Sanofi licencie 400 personnes en recherche et développement, Valvena a quitté le territoire et prospère, aidée par des capitaux anglais. Où est la France ? » L'histoire va-t-elle malheureusement se répéter ? Cette carte d'identité numérique, qui se dit « sécuritaire », n'est qu'un miroir aux alouettes et ne tiendra pas sur le long terme. Les techniques retenues sont anciennes et datent en moyenne de dix ans. Or la durée de vie d'une carte d'identité est justement de dix ans : cherchez l'erreur ! Ainsi, l'encre suisse qui a été retenue a plus de trente ans d'ancienneté. On peut l'acheter sur la plateforme de vente en ligne chinoise AliExpress pour 177 euros.

comment l'Imprimerie nationale, garante de cette carte d'identité, peut-elle préférer des technologies étrangères et dépassées à nos technologies françaises innovantes, alors que l'on sait que ces cartes peuvent être contrefaites ? Pouvez-vous, monsieur le ministre nous rassurer à double titre : premièrement, sur le fait que toutes les garanties sont bien prises en matière de compétitivité technologique et économique ; deuxièmement, au-delà de ce sujet précis, sur la façon de mieux prendre en compte les start-up françaises dans la commande publique.

Nos paysans ne peuvent plus se contenter de belles promesses ; il leur faut aussi des actes, à la vitesse de vos déplacements. Nos agriculteurs sont à genoux, sans aucune trésorerie,

Vous avez annoncé que l'État allait débloquer des enveloppes exceptionnelles. C'est indispensable, mais c'est insuffisant pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu. Il faut réfléchir à des mesures structurelles et pérennes, afin de prémunir notre agriculture de ces aléas climatiques de plus en plus fréquents, notamment par le biais de la création d'aides à l'adaptation des exploitations au changement climatique, afin de les faire évoluer vers des cultures moins fragiles ou moins précoces. Il faut également entamer un travail de fond sur les processus assurantiels. Concrètement, sous quel Concrètement, sous quel délai les sinistrés pourront-ils bénéficier des aides promises ? Au-delà de ces situations de détresse, quelles mesures envisagez-vous pour garantir l'avenir de ce secteur ?

La bataille pour l'or bleu et les déchets se termine donc par un compromis « de bon sens », selon certains. Cet accord préserverait l'intégrité de Suez sur le plan social et industriel tout en lui permettant de se recentrer sur les activités françaises de l'eau et des déchets. Le nouveau Suez devrait être détenu par des actionnaires sans doute « majoritairement français », avec les fonds Meridiam, Ardian et l'américain GIP, qui doivent s'engager pour quatre ans à maintenir l'emploi et les acquis sociaux. Bref, tout va bien ! Le Gouvernement se félicite du transfert de la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement, de la gestion d'une ressource naturelle fondamentale, au profit d'acteurs qui n'ont ni le savoir-faire ni les capacités financières, avec des engagements de court terme sur l'emploi et les acquis sociaux. Qu'en sera-t-il dans quatre ans ? Et quel sera l'avenir de la recherche et du développement, filière d'excellence de Suez ? Vous acceptez une nouvelle désorganisation industrielle et laissez se mettre en place un monopole privé dans un secteur aussi essentiel, sans vous inquiéter des conséquences pour les collectivités locales

Nous allons assister à la création d'un leader mondial autour de Veolia, avec 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'eau et les déchets. Nous allons voir naître un nouveau Suez- pour reprendre votre expression dans l'eau et les déchets au niveau français, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 7 milliards d'euros et, comme vous l'avez vous-même souligné, des investisseurs de long terme, majoritairement français, ce qui est gage de sécurité pour l'ensemble de l'entreprise et des emplois. Le groupe Veolia a réitéré sa volonté de tenir l'intégralité des engagements sociaux qui avaient été pris. Nous veillerons de manière extrêmement attentive à ce que ces engagements soient tenus. Cet accord consacre aussi

Monsieur le ministre, ce n'est pas un accord amiable : c'est une trahison ! Une trahison de l'intersyndicale de Suez, tenue totalement à l'écart des négociations trahison de l'État, qui n'a plus prise sur ces entreprises absolument stratégiques. Il y a pourtant urgence à garantir un droit effectif à l'eau, comme nous le proposerons demain dans cet hémicycle. Il faut aider les collectivités qui veulent rétablir la gestion de l'eau en régie et rendre les premiers litres gratuits. il faut maintenir l'emploi et les filières d'excellence dans notre pays, ce que cette fusion fragilise.

Dans le roman de Victor Hugo, l'archidiacre Frollo refuse de prêter de l'argent à son frère cadet, qu'il aime pourtant comme un fils, de peur qu'il l'utilise à mauvais escient.

la difficulté de la mission de l'établissement public et je sais aussi l'efficacité du dispositif. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la transparence ?

Monsieur le sénateur Bargeton, vous soulignez à juste titre l'émotion considérable qui nous a tous voilà deux ans, lors de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Cette émotion a été considérable, en France et dans le monde entier. Elle s'est concrétisée par une souscription publique qui a réuni 830 millions d'euros de dons, une somme totalement inédite. Je suis bien évidemment garante de la bonne utilisation des fonds et de leur transparence. Dans ce cadre, la Cour des comptes a émis un certain nombre de préconisations que nous avons suivies, et même anticipées,

Aujourd'hui, la solidarité nationale s'impose. Les réponses qui seront apportées ne devront laisser aucun agriculteur sur le côté. Face à ce gel généralisé, répondre à l'urgence sur le terrain doit être notre priorité. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher d'apporter des solutions pérennes pour éviter ces catastrophes économiques et humaines. Du fait du dérèglement climatique, ces aléas- gel, grêle, sécheresse, excès d'eau ... -sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, alors que seuls 30 % de la ferme France sont assurés. Monsieur le ministre, le temps est venu de repenser l'assurance récolte sur l'ensemble du territoire, et bien entendu de la rendre accessible à tous nos agriculteurs. Pour cela, il nous faut abaisser la franchise à 20 % et relever le niveau de subvention à 70 %, comme le prévoit le règlement européen Omnibus. D'autres propositions innovantes pourraient être mises sur la table. Je pense, par exemple, au pool de réassurances pratiqué en Espagne, qui permet de mutualiser les risques. Dans son allocution du 12 mars 2020, le Président de la République déclarait que déléguer notre alimentation à d'autres était une folie. Oui, protéger notre agriculture, c'est protéger notre souveraineté ! C'est bien là le rôle et la place de l'État. Je suis persuadé que, comme pour les catastrophes naturelles, les Français sont prêts à faire preuve de solidarité pour défendre notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. En ce sens, monsieur le ministre,

accompagner nos agriculteurs face à des aléas climatiques dont ils n'ont pas la responsabilité, mais dont ils sont les premières victimes ? Permettez-moi de rebondir, monsieur le sénateur,

les efforts mis en oeuvre par les agriculteurs n'ont pas suffi. La viticulture, mais aussi l'arboriculture, le maraîchage et les grandes cultures ont été dévastés. Des parcelles épargnées par les plus virulents épisodes de 2017 et de 1991 ont gelé en totalité.

ses paysages, mais aussi les fondements de son économie. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, ce sont non pas des mesures de relance, mais un véritable plan de sauvetage de la filière vitivinicole française qu'il vous faut mettre en place.

L'an dernier, j'avais présenté une proposition de résolution avec mes collègues Yvon Collin et Henri Cabanel. Vous devez nous aider à finaliser ce travail face à l'Europe et face aux assureurs. Pour rendre ce dispositif incontournable, il faut baisser le seuil de déclenchement des pertes de rendement, augmenter le taux de subvention et, surtout, revoir la méthode de calcul de la base assurable fixée sur une moyenne olympique par l'Europe. Voilà plus d'un an, l'Association nationale des élus de la vigne et du vin était sur le point d'organiser un Grenelle de la viticulture, pour établir une stratégie globale de filière en réunion interministérielle. Nous souhaitons le relancer et comptons sur votre soutien, monsieur le ministre. L'urgence est réelle ! Rassurez la filière sur le long terme. La parole

Monsieur le ministre, vous avez parfaitement décrit la dimension historique de la catastrophe agricole provoquée par le gel. En Ardèche, où vous vous êtes rendu avec le Premier ministre, la vigne, les arbres fruitiers et, en particulier, les cerisiers et les abricotiers accusent des pertes allant de 90 % à 100 %. Vous l'avez déclaré : « À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. » Soit ! Le Gouvernement doit donc organiser la solidarité nationale, en s'écartant du schéma classique que nos agriculteurs ne connaissent que trop et qui se caractérise par son cortège de lenteurs, de tracasseries et d'injustices. La France, qui, en temps de crise, sait sauvegarder ses banques en quelques jours ou nationaliser ses entreprises stratégiques, peut et doit sauver du désastre ceux qui la nourrissent. C'est pourquoi je souhaite vous interroger sur le caractère exceptionnel de l'action de l'État concernant l'inclusion de toutes les filières frappées, notamment la viticulture, sur la simplicité des démarches que les exploitants devront effectuer et, surtout, sur la rapidité des indemnisations. Monsieur le ministre, les trésoreries des exploitations ont été très éprouvées par la sécheresse de 2020, les taxes américaines sur le vin et la crise du covid. Allez-vous, pour la survie de nos filières, engager cette course contre leur mort économique ?

de l'autonomie. De nombreux professionnels nous alertent sur les souffrances psychologiques et psychiques éprouvées par un grand nombre d'enfants et d'adolescents dans notre pays. Ces jeunes subissent en effet de plein fouet les effets directs et indirects de la crise sanitaire, ceux-ci s'ajoutant parfois à un contexte familial déjà difficile ou qui s'est détérioré à la suite des périodes de confinement. Face à cette situation préoccupante, nous constatons l'impossibilité actuelle de répondre aux nombreuses situations de détresse, faute des moyens suffisants pour faire face à l'augmentation des demandes : centres médico-psychologiques saturés, pénurie de lits d'hospitalisation à temps complet, manque d'effectifs de pédopsychiatres, la liste des carences s'allonge et inquiète. L'ensemble de ces insuffisances structurelles entraîne une discontinuité, voire de graves défaillances dans les prises en charge individuelles, laissant les professionnels sociaux et médico-sociaux bien seuls face à des situations qui nécessitent pourtant un accompagnement renforcé et, surtout, pluridisciplinaire. Madame la ministre, chaque jour, nous voyons de nouvelles formes de souffrances psychiques se développer chez des enfants et adolescents de plus en plus jeunes : violences, addictions, tentatives de suicide ... Le risque de nouveaux passages à l'acte ne cesse de s'amplifier. Quelles mesures concrètes et urgentes le Gouvernement compte-t-il appliquer pour parer à cette détresse grandissante de nos jeunes, en particulier pour les plus fragiles d'entre eux ? La parole de l'autonomie. Monsieur le sénateur Jean-Luc Fichet, la psychiatrie infantile, vous le savez, souffre de difficultés structurelles bien connues depuis de nombreuses années. ni de cette mandature ni même de la crise sanitaire. Les départs à la retraite des effectifs médicaux spécialisés et l'augmentation sensible de la demande de soins ont suscité des situations de saturation, exacerbées par la crise sanitaire en cours. C'est un enjeu qui préoccupe pleinement le Gouvernement. Si peu de données consolidées existent, nombre de signes nous alertent : troubles du sommeil, dépressions et tentatives de suicide, que vous évoquiez. Les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés autour de Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, et d'Adrien Taquet, secrétaire d'État,

a été nommée au Conseil scientifique pour assurer la prise en compte de l'impact des mesures sur les enfants. Cette après-midi, le chef de l'État se rendra à Reims, accompagné du ministre Olivier Véran et du secrétaire

permettra également de revenir sur les chantiers en cours pour répondre à l'urgence, mais aussi, de manière structurelle, aux attentes de ce secteur clé.

Monsieur le Premier ministre, je veux vous interpeller sur le fonctionnement actuel du conseil des ministres. C'est l'organe constitutionnel de la délibération gouvernementale. Or, en ces temps de crise sanitaire, il est non plus réuni à l'Élysée, mais remplacé par une réunion à distance, ce qui pose trois problèmes. d'un problème institutionnel, la collégialité de la délibération gouvernementale n'étant pas assurée dans les formes constitutionnelles. Cela crée pour l'avenir un précédent préoccupant.

depuis 2003 la loi qui n'a pas été délibérée correctement en conseil des ministres avant son examen par le Parlement. Dans ces conditions, monsieur le Premier ministre, allez-vous demander au Président de la République de rétablir le fonctionnement normal du conseil des ministres ?

de membres du Gouvernement assistant « en présentiel », comme on dit, au conseil des ministres a en effet été limité depuis le début de la crise.

La notion de délibération renvoie à la possibilité d'un échange de vues et de prises de parole des membres du conseil des ministres. Pour considérer que le conseil des ministres a été valablement réuni, il convient donc d'examiner non pas s'il a donné lieu à une réunion physique de ses membres, mais si des modalités d'organisation lui ont effectivement permis de délibérer. atteste, c'est bien ce qui se passe. À cet effet, il est fait recours à un dispositif de visioconférence, porté par un système sécurisé de niveau confidentiel défense, conçu et opéré par l'État,

J'apprécie, monsieur le Premier ministre, que vous vous soyez donné la peine de me répondre personnellement. Toutefois, je voudrais vous dire, avec la plus grande solennité, que l'argument sanitaire ne tient pas. D'ailleurs, vous ne seriez pas ici pour nous répondre si nous appliquions la même règle que celle que vous prétendez voir s'imposer pour le conseil des ministres. Pourtant, votre sécurité sanitaire, comme celle des membres du Gouvernement, est assurée aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. dispose à l'évidence de salles qui ont la dimension nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire des ministres. Vous ne devez plus prendre le risque de dégrader,

La liberté des autres étend la mienne à l'infini. » En Birmanie, Aung San Suu Kyi est sous le coup de nouvelles poursuites pénales. Depuis le coup d'État qui l'a chassée du pouvoir le 1 février dernier, la situation ne cesse de se dégrader. Plus de 700 civils ont été tués par une junte mortifère et de plus en plus organisée. Un culte impressionnant de la personnalité se renforce autour du chef, avec des défilés militaires dignes des plus grands régimes autoritaires, ce qui conforte l'armée dans son action et fait croître la répression sanglante des manifestations. Désormais, les militaires n'hésitent plus à tuer jeunes ou moins jeunes, pacifistes ou militants. Ces hommes et ces femmes qui luttent héroïquement pour leur liberté sont abattus par des, preuve de plus, s'il en fallait, de cette répression criminelle et intolérable. Ce week-end encore, 82 personnes ont perdu la vie. L'ambassadrice de l'ONU, venue spécialement, n'a pas été autorisée à entrer dans le pays. La communauté internationale peine une nouvelle fois à s'affirmer, en raison des vétos russes et chinois. Aung San Suu Kyi est détenue dans un lieu tenu secret. Six chefs d'accusation sont retenus contre elle, dont celui de corruption, qui pourrait l'empêcher d'exercer toute fonction politique. face à ce silence total et assourdissant, la France, pays des droits de l'homme, ne peut pas rester sans rien dire. La non-reconnaissance de la junte par l'État français n'est plus suffisante. L'Union européenne doit aussi s'imposer et répondre d'une seule voix. Les vétos de l'ONU ne sont pas des raisons acceptables pour laisser de tels crimes impunis ; nous devons agir. Quelles sanctions allez-vous prendre pour enrayer la tragédie endurée par les Birmans, désespérément seuls face à leurs tortionnaires ?

démarches réalisées au niveau des Nations unies, puisque nous avons soutenu fortement la consultation menée la semaine dernière avec des représentants de l'opposition.

le biais d'un courrier, et cela, de manière purement fortuite, au lendemain même des dépôts des listes pour les élections consulaires du mois de mai

communication institutionnelle et communication politique, ... Comme souvent ! ... en utilisant, de surcroît, une base de données exclusivement réservée à des finalités administratives, contrairement à la liste électorale consulaire. C'est moralement condamnable et politiquement déloyal. Moralement condamnable, car l'utilisation d'un registre à des fins électoralistes constitue une violation par le Président de la République lui-même d'un principe essentiel en démocratie, à savoir l'égalité de traitement entre les candidats. Politiquement déloyal, parce que cette correspondance, parsemée d'autosatisfaction, s'apparente à un plaidoyer en faveur des candidats La pour les futures élections. Monsieur le secrétaire d'État, comment pouvez-vous justifier l'utilisation de moyens étatiques à des fins de propagande, à un moment électoral clé pour les Français établis hors de France ?

oui, le Président de la République est particulièrement attentif à la situation des Français établis hors de France ! Oui, le Président de la République les considère comme des Français à part entière, et non comme des Français à part tout court. ! Permettez-moi de le relever, dans ce courrier, le Président de la République salue l'action de l'ensemble des élus des Français de l'étranger, les élus locaux, mais également les parlementaires qui siègent ici.

En juillet 2020, les conclusions du Ségur de la santé actaient une revalorisation salariale pour les agents hospitaliers, laissant de côté nombre d'agents exerçant pourtant les mêmes métiers dans les établissements du secteur social et médico-social. Les oubliés du Ségur ont dû batailler pendant de longs mois pour faire entendre cette injustice et arracher une juste reconnaissance et une revalorisation méritée de leur rémunération. Ils et elles ont eu raison de se mobiliser, notamment les professionnels du soin à domicile, dont nous souhaitons le développement. Vos annonces intervenues lundi dernier, madame la ministre, laissent à penser que cet oubli serait réparé. S'il faut se satisfaire que votre gouvernement s'engage enfin à ouvrir cette revalorisation au personnel paramédical sans distinction du statut de leur employeur, et si nous saluons l'extension de la revalorisation au personnel éducatif du secteur du handicap, de nombreuses incertitudes demeurent. Quelle revalorisation prévoyez-vous pour les nouveaux oubliés : les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, qui s'acquittent des mêmes tâches éducatives, sanitaires ou sociales, les travailleurs sociaux des foyers d'accueil médicalisés des instituts médico-éducatifs, pourtant aussi essentiels aux personnes en situation de handicap, les psychologues hospitaliers, les sages-femmes- profession médicale toujours sous-valorisée -et les infirmiers anesthésistes Madame la ministre, envisagez-vous sérieusement de financer ces promesses, alors que vous repoussez encore la discussion parlementaire sur les moyens accordés au grand âge et à l'autonomie ? Allez-vous envoyer la facture aux départements ?

Les Républicains. Madame la secrétaire d'État, plusieurs de mes collègues sont intervenus la semaine dernière sur l'aide publique accordée à Air France. Je souhaite pour ma part aujourd'hui vous interroger sur le choix du repreneur des dix-huit créneaux que la compagnie devra céder à Orly, pour respecter les règles de concurrence. M. Djebbari a assuré la semaine dernière que le Gouvernement éviterait tout dumping social ou fiscal, mais rien n'a été dit sur les critères environnementaux. Rien n'empêche des compagnies de candidater.

Ces avions sont plus polluants et plus bruyants. Il ne faudrait pas, d'un côté, imposer à la société Air France d'être plus attentive à l'environnement et la forcer à innover, ce qui est une des conditions de l'aide publique, et, de l'autre, permettre à ses concurrents, ou non, d'opérer à sa place sur notre territoire avec des avions plus polluants. Plusieurs villes du Val-de-Marne, dont Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Ablons ou Orly se plaignent depuis des années des pollutions liées à l'aéroport. Sachez que ni les élus, ni les parlementaires, ni les riverains n'accepteront que la réattribution des créneaux aggrave la situation. Le ministère des transports siégeant au conseil d'administration de l'Association pour la coordination des horaires, pouvez-vous m'assurer que le Gouvernement veillera à ce que ce choix respecte les critères environnementaux essentiels ?

nous avons veillé à ce que cela ne fragilise pas Air France et ne compromette pas sa réorganisation, notamment le développement de l'activité de Transavia. Cet accord prévoit que le bénéficiaire des créneaux qui seront mis à disposition, de façon pérenne, par Air France ses avions et les équipages qui leur sont liés à Orly et respecte pleinement le droit du travail européen et national. Les autorités françaises se sont d'ailleurs attachées à prévoir un mécanisme de contrôle qui permettra de sanctionner les éventuels manquements à cette

lors de ces négociations avec la Commission, nous avons été très vigilants pour que la solution retenue ne provoque en aucun cas une aggravation des nuisances sonores et environnementales subies par les riverains de l'aéroport et pour que le plafonnement des mouvements et le couvre-feu demeurent inchangés.

la santé, chargée de l'autonomie. Elle porte sur la rémunération des professionnels de santé actuellement engagés dans la campagne de vaccination. Tout travail mérite salaire. Il aura pourtant fallu trois mois pour que, enfin, le travail du personnel de santé, notamment des retraités intervenant dans les centres de vaccination covid, soit reconnu.

De nombreuses questions restent donc sans réponse : les cotisations sociales s'appliquent-elles pour les retraités ? Comment procédez-vous au remboursement des structures qui ont avancé la rémunération de leur personnel ? Quelle plateforme efficace sur le long terme Enfin, que comptez-vous faire, madame la ministre, pour accélérer la rémunération des personnels de santé retraités engagés dans la campagne de vaccination covid ? La parole Madame la sénatrice Jocelyne Guidez, votre question est double. Je tâcherai donc de répondre à chacune des dimensions que vous évoquez. La mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé retraités est à l'image de la solidarité qui s'est développée dans notre pays de manière spontanée. Je tiens à rendre hommage à ce dévouement et à cette mobilisation, qui se

de mettre en oeuvre rapidement les modalités les plus efficaces et les plus adaptées pour verser leurs salaires à ces professionnels. Sachez que c'est désormais chose faite, puisque leur paiement direct est assuré depuis le 1 avril 2021, y compris

intervenant à titre exclusif, ainsi que les professionnels exerçant sur des lieux non conventionnés avec leur centre habituel de rattachement. Nous nous sommes donc assurés qu'une solution

pour limiter le plus possible le type de situation que vous évoquez. Ces difficultés devraient disparaître progressivement dans les prochaines semaines. La parole

en application de l'article 50-1 de la Constitution, relative à l'organisation des prochaines élections départementales et régionales. Cette séance s'organisera en

Monsieur le président,

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote, en application de l'article 50-1

ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le 1 avril dernier, je suis venu présenter devant vous la situation sanitaire de notre pays, marquée, vous le savez, par une troisième vague d'un nouveau variant prédominant, ainsi que les mesures de lutte contre l'épidémie que l'évolution de cette situation sanitaire nécessaires. Voilà donc plus de dix jours que ces dispositions sont entrées en vigueur sur l'ensemble du territoire. Elles commencent à produire leurs résultats en termes d'incidence, même si c'est de manière hétérogène selon les régions, mais pas encore en termes de pression hospitalière. Plus que jamais, la communauté des soignants se mobilise pour faire face à cette pression, avec la compétence et le courage qui lui valent plus que jamais notre reconnaissance et notre soutien. C'est dans ce contexte très particulier que j'ai évoqué devant la Haute Assemblée le calendrier des prochaines élections départementales et régionales, fixées les 13 et 20 juin prochain, que les questions soulevées par le conseil scientifique dans le rapport qu'il nous a remis, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 22 février 2021, relatif aux conditions de leur organisation.

Elle a toujours été constante et repose sur un principe très simple : celui du maintien- c'est la règle -, parce que l'élection est un moment majeur de la démocratie et, de surcroît, les élections en question ont déjà dû être reportées. reportées. Seules des considérations sanitaires- c'est l'exception -pourraient nous conduire à déroger à ce principe ou à en aménager l'organisation, comme l'a démontré, du reste, l'expérience difficile des élections municipales de l'année dernière. Privilégier l'hypothèse du maintien, c'est aussi identifier clairement et lucidement les difficultés que sa mise en oeuvre peut soulever. Ces difficultés tiennent évidemment aux contraintes et aux incertitudes que la situation sanitaire peut faire peser sur notre vie collective dans les prochains mois. Elles tiennent plus particulièrement aux recommandations très précises que le conseil scientifique a formulées, qu'il s'agisse des conditions de déroulement de la campagne

Elles tiennent enfin au fait que ces élections cumuleront deux scrutins- cela les distingue des municipales de 2020 -, organisés le même jour, ce qui exige de doubler le nombre de bureaux de vote, donc de mobiliser deux fois plus de présidents et d'assesseurs. Faut-il rappeler, par ailleurs, qu'après l'avis du conseil scientifique, nous avons nous avons renforcé, à compter du 4 avril et pour une période de quatre semaines, les mesures dites « de freinage », et que ceci n'est évidemment pas sans effet sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, s'agissant notamment de la précampagne électorale

J'ai saisi les présidents des assemblées, les présidentes et présidents des groupes parlementaires, les responsables des partis politiques représentés au Parlement et les responsables des associations d'élus locaux.

Une assez large majorité de ces contributions- 25, pour être précis -a exprimé une position favorable au maintien des dates prévues, 11 n'ont pas pris

d'autres ont souligné les difficultés qui pouvaient se poser et quelques-unes étaient accompagnées de propositions précises de nature à y remédier. L'importance du sujet et les conditions précises fixées par le conseil scientifique m'ont par ailleurs convaincu de procéder à une consultation directe des maires.

dans la mesure où le principal effort et la responsabilité de l'organisation de ces scrutins pèseront nécessairement sur les maires. Je tiens d'ailleurs à les remercier devant vous, dans cette assemblée dont ils sont les grands électeurs,

Celles-ci ne surprendront personne, tant ces élus montrent depuis le début de cette crise leur disponibilité et leur engagement, en tous points exemplaires, au service de notre pays. Leurs préconisations, leurs très nombreuses contributions, comme les interrogations qu'ils ont soulevées, enrichissent considérablement l'information tant du Gouvernement que du Parlement, notamment dans le cadre du présent débat. Cela n'a rien de surprenant, puisqu'elles émanent de celles et ceux dont c'est précisément la charge et la mission que d'assurer l'organisation matérielle des opérations de vote. Les élus municipaux intervenant dans le processus électoral comme agents de l'État,

et, surtout, au vu de leurs légitimes inquiétudes, s'il ne les accompagnait pas au plus près dans l'organisation de ces opérations dans le contexte très particulier que nous connaissons. Contrairement à ce que certains commentaires ont parfois laissé entendre, cette consultation- à l'indiquer de manière très solennelle -n'était dirigée contre personne et certainement pas contre les associations d'élus, pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Je sais d'ailleurs que le Sénat lui-même a pour habitude, et cela me semble bien normal, de consulter directement les élus locaux, deux consultations de ce type étant en cours. C'est une bonne méthode. Il s'agissait tout simplement, je le répète, de compléter utilement les réponses des associations, en donnant une dimension très concrète et opérationnelle aux questions de principe soulevées à bon droit par les contributions des grandes associations d'élus. Vous connaissez le résultat de cette consultation : 56 % des maires se sont prononcés en faveur du maintien, 40 % en faveur du report et 4 % n'ont pas souhaité prendre position. Ces résultats montrent à eux seuls combien le sujet est complexe-

sont exprimées. J'en viens enfin au rendez-vous que je vous avais proposé et qui nous réunit aujourd'hui sous la forme de ce débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution et du vote qui le conclura. il faut que, en toute transparence, chacun puisse s'exprimer et s'engager au regard des enjeux qui sont sur la table, puisqu'il s'agit de concilier les deux principes de portée constitutionnelle que sont la liberté du suffrage et la protection sanitaire de nos concitoyens. Ce débat et ce vote, je vous propose donc de les organiser sur la proposition, confirmant l'orientation dont je vous avais déjà fait part, de maintenir au mois de juin les élections régionales et départementales et d'assortir ce maintien de conditions très précises, tenant à la campagne comme au vote, conditions que je développerai dans un instant. Cette position est celle qui apparaît au Gouvernement comme prenant le mieux en compte à la fois l'avis du conseil scientifique du 29 mars dernier et le résultat de l'ensemble des consultations que nous avons conduites depuis lors et que je viens de vous rappeler. S'agissant en premier lieu de la campagne électorale, celle-ci devra donc être adaptée. Comme l'a rappelé le conseil scientifique, c'est elle qui est de nature à entraîner une multiplication des occasions de contacts physiques, donc d'accroître les risques sanitaires. Cette campagne sera donc différente ; du reste, la quasi-totalité des forces politiques consultées en convient. Ainsi, nous encouragerons l'usage des outils de campagne dématérialisés. Le ministère de l'intérieur mettra en place, comme pour les dernières municipales, un site internet permettant aux électeurs de disposer de l'ensemble des professions de foi des candidats aux deux élections. Un débat télévisé, également diffusé à la radio, sera organisé entre les candidats aux élections régionales, avant chacun des deux tours de scrutin. Le Gouvernement, de son côté, lancera une grande campagne de sensibilisation au vote, ainsi qu'une campagne d'information sur les compétences des conseils régionaux et départementaux. Le conseil scientifique recommande, en outre, l'interdiction des meetings physiques et des réunions publiques, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans la période de restrictions sanitaires que nous connaissons actuellement, une telle règle me paraît justifiée. Je souhaite toutefois qu'elle puisse être réévaluée, dès que l'amélioration de la situation sanitaire nous permettra d'envisager la reprise progressive de certaines activités et l'ouverture de quelques établissements recevant du public.

Ces règles seront donc aménagées sans délai, afin d'autoriser les déplacements des candidats dans le ressort de la circonscription électorale, ainsi que des militants qui les accompagnent, sur la base d'une attestation du candidat ou, à défaut, de son mandataire financier. Pour prendre en compte l'allongement de la campagne, nous allons, comme pour les élections municipales de juin 2020, augmenter la durée des prêts accordés par les personnes physiques.

il nous appartient de prendre toute disposition utile afin d'assurer la sécurité sanitaire des personnes concourant aux opérations de vote et, plus généralement, de tous les électeurs. Comme pour le second tour des municipales, en juin dernier, un protocole sanitaire sera défini de façon à garantir le respect des gestes barrières et la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Le recours au vote par procuration sera de nouveau facilité : la loi du 22 février 2021 offre à chaque électeur la possibilité de disposer de deux procurations.

permet d'établir une procuration de façon presque totalement dématérialisée. Le conseil scientifique recommande également la vaccination ou, à défaut, le dépistage de l'ensemble des membres des bureaux de vote.

été protégée, et nous espérons faire mieux ! C'est pourquoi le Gouvernement propose de mettre en place un dispositif spécifique : trois semaines avant le premier tour, les communes seront invitées à faire connaître la liste des personnes non vaccinées, membres des bureaux de vote, et des fonctionnaires mobilisés le jour du scrutin, afin qu'une vaccination puisse leur être proposée. Le conseil scientifique prévoit que, à défaut de vaccin, les membres des bureaux de vote devront réaliser un test.

les communes de lots d'autotests leur permettant de tester, le jour du scrutin, tous les participants aux opérations de vote qui n'auraient pas eu d'autres solutions. Afin de limiter les concentrations de flux d'électeurs, et comme de nombreuses forces politiques l'ont proposé, les préfets seront invités à étendre les horaires des bureaux de vote de huit heures à vingt heures, dans toutes les communes où, après échange avec

des mesures seront prises pour préciser les textes relatifs à la mutualisation des équipements et de certaines fonctions des membres des bureaux de vote. Afin de limiter le nombre de personnes mobilisées par les opérations de dépouillement,

C'est pourquoi les préfets et les sous-préfets seront chargés de les accompagner de manière individualisée, dans la préparation et l'organisation des scrutins. L'État ne laissera pas les maires des petites communes livrés à eux-mêmes : dès lors, l'accompagnement préfectoral commencera très prochainement, en vue d'identifier le plus précocement possible les difficultés prévisibles et d'y apporter des solutions adaptées. Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs des mesures que je viens de vous présenter relèvent de la loi. Les dispositions correspondantes seront intégrées à un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui sera présenté d'ici à la fin du mois d'avril en conseil des ministres. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà le cadre général que je soumets à votre approbation. Sa déclinaison opérationnelle supposera l'adoption d'actes juridiques et matériels nombreux et importants. devront être adoptés dans des délais très rapprochés- c'est un défi ! Nous devrons être en mesure de répondre à de nombreuses conditions, d'adopter de nouvelles dispositions législatives et réglementaires, de déployer des moyens d'information novateurs et inédits, d'accompagner les mairies dans l'organisation matérielle du scrutin. En outre, et c'est essentiel, nous devrons compter sur le bon avancement de la campagne de vaccination. Les semaines qui nous séparent du scrutin ne seront pas de trop pour relever ce défi collectif. C'est pourquoi, pour nous donner le temps utile, nous avons décidé de décaler d'une semaine la date des élections. effet, une semaine de plus, cela représente deux à trois millions d'électeurs vaccinés supplémentaires.

À cet effet, un comité de suivi permanent, présidé par Jean-Denis Combrexelle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et animé par le ministère de l'intérieur, sera constitué. Il associera les membres des partis politiques représentés au Parlement, les groupes parlementaires et les associations d'élus. Il examinera, au fil de l'eau, si vous me permettez cette expression, toutes les questions juridiques et organisationnelles de la campagne et du scrutin. J'ajoute, pour votre complète information, qu'un préfet sera désigné pour piloter les sujets à caractère logistique, afin de soutenir les maires dans l'organisation du scrutin, y compris au regard des enjeux liés au dépistage et à la vaccination. Le ministre de l'intérieur, dont je veux saluer l'implication à mes côtés, sera chargé, au nom du Gouvernement, de mettre en oeuvre l'ensemble des orientations que je viens de vous exposer.

Monsieur le président, Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, il y a un an, notre pays entrait dans une crise sanitaire sans précédent. crise n'est naturellement pas terminée, nous ne le savons que trop. Elle a provoqué des drames dans les familles

on commençait alors à parler du vaccin et, au début du mois de janvier, revenait dans le débat la question des élections.

en accepta le principe. Vous recueillîtes, monsieur le Premier ministre, l'avis favorable de toutes les organisations d'élus locaux, et nous décidâmes ensemble, en février dernier, que ces élections auraient lieu en juin.

Eh bien non, les maires répondirent et libérèrent le Gouvernement, en affirmant massivement qu'ils voulaient ces élections, quand bien même les associations avaient déjà donné un avis positif. Je vous accorde, monsieur le Premier ministre, que la majorité n'est pas extrêmement large, mais elle est tout de même suffisamment nette pour considérer que ces élections puissent avoir lieu. Et vous avez décidé, à juste raison, de maintenir les élections et de venir devant nous le confirmer.

texte nous engage, et nous n'avons pas changé. En revanche, vous avez sollicité le Parlement, et nous vous en remercions, sur les conditions dans lesquelles cette élection pourrait se dérouler. Cette consultation a permis à la commission des lois, que j'ai l'honneur de présider, de débattre la semaine dernière et de formuler un certain nombre de propositions, que nous avons transmises au président du Sénat. Il vous les a lui-même adressées le 8 avril dernier.

Leurs relations sociales sont contraintes par les restrictions sanitaires et leurs proches n'ont jamais été si loin. Ces chambardements ont dessiné, pour chacun de nous, un nouveau quotidien dans tous les aspects de nos vies. La vie démocratique, qui n'est jamais qu'un seul de ces aspects, a profondément évolué au gré de la situation sanitaire. Il est vrai que, en ce moment, la vie démocratique ne ressemble pas à ce qu'elle était avant la pandémie. gré, elle suit son cours. Il faut dire que tout avait commencé sous de sombres auspices, par l'annonce du premier confinement le 14 mars 2020, à la veille des élections municipales. On connaît la suite : maintien du premier tour malgré la sidération et l'inquiétude. Les élus locaux, les assesseurs et les présidents de bureaux de vote ont été fidèles au poste : leur engagement exemplaire a permis la bonne tenue de ce scrutin, si essentiel à la démocratie locale. Depuis lors, presque toutes les élections ont pu se tenir, malgré des aménagements substantiels. Force est de constater que ces aménagements, s'ils ont profondément changé le visage des élections- notamment pour les municipales, dont le second tour s'est tenu plusieurs mois après le premier -, n'ont finalement pas entamé la légitimité des élus, fort au contraire. Je pense, bien évidemment, aux dernières élections sénatoriales- j'en suis issue -, qui ont concerné la moitié d'entre nous. Je pense également aux renouvellements des conseils intercommunaux ou encore aux élections professionnelles, qui concourent à la vitalité du dialogue social. Au Parlement, comme dans tous les conseils communaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux, la vie démocratique s'est adaptée. Qui, au Sénat, pourrait affirmer le contraire ? Comme partout en France, la Haute Assemblée a dû composer avec les contraintes sanitaires, tandis que nos méthodes de travail ont évolué. Nous avons pleinement rempli nos fonctions de parlementaires, même si nous l'avons fait de façon inédite et parfois insolite. Depuis mars 2020, presque toutes les élections ont donc pu se tenir, exception faite des élections départementales et régionales, nous avons déjà voté un premier report à cause de la deuxième vague. Il s'agit, aujourd'hui, de savoir s'il faut opter pour un nouveau report face à une nouvelle vague. Admettons, tout d'abord, qu'il est plus que légitime de se poser la question. Par rapport à cet hiver, la situation a largement évolué. D'une part, la campagne de vaccination, notamment compte tenu de l'accélération récente qu'elle a connue, nous permet d'envisager une période d'accalmie, avec le retour des beaux jours. D'autre part, la propagation des variants, entre autres complications, nous incite à la prudence. En tout état de cause, deux choses sont à ce stade certaines. Tout d'abord, personne, ici, ne peut garantir que la situation sera nettement meilleure en juin prochain qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si de nombreux indicateurs nous permettent légitimement de l'espérer.

Nous devons donc nous rendre à l'évidence : au cours des prochains mois, la situation demeurera placée sous le signe de l'incertitude. Toutefois, plusieurs éléments nous permettent d'envisager plus sereinement la bonne tenue d'un scrutin en juin prochain. J'identifie au moins trois arguments dans ce sens. Le premier, c'est que nous avons acquis, depuis les élections municipales, une précieuse expérience en matière d'organisation de scrutins par temps d'épidémie. De manière plus générale, nous avons appris à vivre avec le virus. Nous nous sommes équipés pour nous protéger et avons intégré les gestes barrières. En somme, nous avons de quoi aborder plus sereinement la tenue des prochains scrutins. Le deuxième argument est l'accélération de la campagne vaccinale. Les chiffres récents sont plutôt encourageants ; il nous faut absolument tenir ce rythme au cours des prochaines semaines, malgré les mauvaises nouvelles liées au déploiement du vaccin Johnson & Johnson. L'objectif des 30 millions de premières doses injectées d'ici à la mi-juin nous laisse envisager une participation plus sereine, notamment de la part de nos concitoyens les plus fragiles. Ces deux premiers arguments ont sans doute emporté la conviction des maires, qui se sont majoritairement exprimés en faveur du maintien du scrutin en juin. Ils compteront, bien sûr, sur le concours de l'État s'agissant des aspects opérationnels de ces prochaines échéances. Tout ce qui pourra être fait en amont pour garantir aux organisateurs les conditions les plus sûres au plan sanitaire mis en oeuvre. Des aménagements de la stratégie vaccinale pourraient d'ailleurs être envisagés, par exemple pour les assesseurs. Notre groupe est ouvert aux discussions sur ce point. Il est bien sûr très important d'écouter l'avis des maires, qui seront concernés au premier chef, même si la décision échoit à l'État. Nombre d'entre nous auraient préféré que la consultation se déroule dans de meilleures conditions, mais l'essentiel est que le Gouvernement puisse prendre une décision en connaissance de cause. Le troisième et dernier argument, c'est que nous pouvons apprendre des nombreux autres pays qui ont fait face à des situations à bien des égards comparables et qui sont, malgré tout, parvenus à respecter leur calendrier électoral. Je pense, bien sûr, aux élections présidentielles aux États-Unis, en novembre dernier. Je pense aussi à nos voisins européens, qui se sont rendus aux urnes et ont trouvé des solutions pour adapter la tenue des scrutins. La flexibilité et l'innovation ont permis de sécuriser les modalités de vote. Le vote par correspondance a pris une place importante, tout comme le vote par anticipation. Dans certaines régions, notamment en Espagne, des plages horaires spécifiques ont été mises en place. De manière moins classique, certains votes se sont déroulés à l'extérieur, par exemple chez nos voisins des Pays-Bas, ou ont été étalés sur plusieurs jours. La démocratie, tout comme les citoyens, fait preuve d'adaptation et d'inventivité, pour dépasser les obstacles auxquels elle est confrontée. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la démocratie est aussi précieuse qu'exigeante. Si elle n'est pas régulièrement exercée, elle court le risque de s'anémier. Très bien ! Ainsi, le maintien des échéances électorales n'a pas à être justifié : il se justifie par la seule nécessité de faire vivre notre démocratie.

considère que, à ce jour, ces raisons ne sont pas réunies. C'est pourquoi nous voterons en faveur du maintien des élections en juin prochain. Le décalage d'une semaine, avec un premier tour fixé au 20 juin

Vous le verrez si vous poursuivez dans la voie que vous esquissez aujourd'hui : on y gagne en sérénité et on dort mieux la nuit. Je vous invite d'ailleurs à passer le message au Président de la République. Le caractère quelque peu expéditif de la consultation nous laisse quelque peu perplexes et nous étonne, pour reprendre vos mots. Nous avons le sentiment, comme trop souvent, que cette consultation est sortie de votre chapeau quelques heures avant son lancement. Pourtant, le rapport du conseil scientifique datait du 29 mars : il y avait matière à laisser une ou deux semaines de battement aux maires. Au-delà du, c'est surtout la question posée aux maires qui interroge interroge : « Les conditions sanitaires préconisées par le conseil scientifique vous semblent-elles réunies pour organiser les deux tours du scrutin en juin ? » Permettez-moi de me faire le porte-parole de nombreux maires de France et de vous retourner la question, monsieur le Premier ministre : les conditions sanitaires vous semblent-elles réunies ? Pensez-vous que l'on aura effectivement vacciné la moitié du pays, dont l'intégralité des personnes à risque, d'ici à la mi-juin ? Pensez-vous que vous serez en mesure de vacciner tous les agents, tous les présidents et tous les assesseurs de bureaux de vote qui en feront la demande ? Pouvez-vous promettre que l'État prendra à sa charge l'ensemble du surcoût des opérations électorales, lequel ne peut pas incomber à des communes déjà exsangues ? Pensez-vous être en mesure de mettre en place suffisamment en amont un protocole sanitaire précis et durable, pour permettre aux maires de s'organiser sans changement de dernière minute ? J'ajoute une dernière question, que les maires se posent moins directement : pensez-vous être en mesure de protéger les candidates et les candidats, comme leurs équipes, ainsi que toutes les personnes qu'ils rencontreront, en favorisant leur accès rapide à la vaccination et en les équipant en autotests ? Voilà autant de réponses dont les maires, comme les parlementaires, auraient aimé disposer pour se prononcer en disposant de toutes les informations nécessaires. Un doute me taraude, monsieur le Premier ministre : qu'attendiez-vous de la réponse des maires ? Qu'elle vous offre un prétexte pour repousser les élections ? Eh oui ! Qu'elle vous permette de vous décharger de la responsabilité de cette décision ? La réponse des maires de France et la forte participation à cette consultation, aussi expresse qu'un sondage sur Twitch, ne nous surprennent pas. L'attachement des maires à notre démocratie L'attachement des maires à notre démocratie ne nous surprend pas davantage : comme nous, ils pensent que, malgré les craintes légitimes, la démocratie ne doit pas être confinée. Aussi, même si nous n'avons pas tous les éléments, même si l'incertitude pèse et continuera de peser sur ce scrutin, nous pensons, comme l'essentiel des forces politiques, que notre démocratie doit vivre avec le virus.

Sauf cataclysme sanitaire, ces élections doivent se tenir. Nous le pensions hier et nous le pensons aujourd'hui. C'est pourquoi nous voterons en faveur de la proposition que vous formulez aujourd'hui. C'est d'autant plus facile que la plupart des modalités d'organisation du scrutin que vous proposez nous conviennent : faciliter faciliter les procurations, même si les propositions adoptées par le Sénat en la matière étaient plus ambitieuses que les vôtres ; élargir les horaires de vote dans toutes les communes où c'est pertinent installer des bureaux en extérieur quand cette organisation est possible ; prévoir une plage horaire privilégiée pour les personnes à risque ; avoir un même scrutateur pour les deux scrutins, comme vous l'avez annoncé ; enfin, créer la possibilité pour les assesseurs et les agents de procéder

J'attire simplement votre attention sur le recrutement des scrutateurs pour le dépouillement. Ce dernier s'annonce complexe : les mêmes précautions de vaccination ou de test seront plus dures à prendre que pour les assesseurs et les agents. C'est bien cette phase du scrutin qui s'annonce la plus délicate. Si, malgré les défis logistiques et sanitaires, l'organisation du scrutin ne semble pas insurmontable, celle de la campagne électorale pose davantage de difficultés. La liberté de déplacement des candidats était nécessaire, vous l'autorisez. Vous proposez une clause de rendez-vous pour les rassemblements en plein air. Très bien ! Toujours est-il que le gros de la campagne sera dématérialisé, et c'est sur ce point qu'il faut concentrer l'effort. Vous prévoyez des campagnes d'informations gouvernementales, un site internet regroupant toute la propagande de tous les candidats à tous les scrutins, des débats sur les chaînes du service public dans toutes les régions : ces mesures représentent un début de solution, mais il faut aller plus loin. Nous vous demandons de doubler l'envoi de la propagande électorale : un premier envoi à un mois du scrutin, un autre, classiquement, la semaine précédant le vote. Nous souhaitons aussi doubler à quatre pages la taille des circulaires dites « professions de foi » : ce sera souvent le seul document que recevront les électeurs, faute de distribution de tracts. Nous vous demandons également d'adresser les instructions nécessaires pour que les panneaux électoraux soient en place dès le début de la campagne officielle, soit le 1juin, afin d'amplifier les possibilités d'affichage. Nous vous invitons également à assouplir la production des clips de campagne et à avancer et élargir leur diffusion sur toutes les antennes locales du service public audiovisuel. Vous envisagez un débat par région sur ces mêmes antennes. C'est un minimum auquel nous vous demandons de veiller. Il n'y a pas de raison en la matière de léser les départements : il est nécessaire d'organiser au moins un Pour cette campagne largement dématérialisée, il faut « mettre le paquet », si j'ose dire, et l'État doit y prendre toute sa part. Dans le flou de la période, peut-être serait-il également opportun que le Gouvernement par une circulaire ce qui relève, dans les moyens d'action et de communication des exécutifs locaux, de l'indispensable lutte contre la pandémie et ce qui participe de l'utilisation de ces moyens à des fins de campagne électorale.

d'éviter qu'une incertitude similaire pèse sur l'élection présidentielle et les élections législatives, ce qui serait démocratiquement catastrophique, allez-vous enfin vous battre pour lever les brevets des vaccins et favoriser leur diffusion en France comme dans le monde, limiter la multiplication des variants ravageurs, et nous permettre de voir, enfin, le bout du tunnel ?

J'entends parfaitement ceux qui affirment que la démocratie ne peut être confinée, que la date d'une élection se décrète en fonction non pas d'une occasion, mais de la loi et du respect de la Constitution.

que la vie démocratique doit respirer, sa respiration sera de type covid, haletante et essoufflée, si la campagne ne peut se dérouler normalement et si les conditions de vote sont trop coercitives.

consulté ! Pourquoi dépassionner le débat et analyser lucidement la situation ne serait-il pas possible ? Repousser les élections de six mois, quand une grande majorité des Français sera vaccinée et qu'une véritable campagne pourra se dérouler, serait, pour les oppositions, une manipulation, une manoeuvre sournoise au service d'intérêts douteux Non ! Mes chers collègues, la majorité ne redoute pas ces élections, pas plus que vous ne redoutez l'élection présidentielle ! Une consultation lucide, sereine représentative doit se dérouler sous trois conditions, par ailleurs très bien décrites par l'un de nos collègues franc-comtois de la majorité sénatoriale. Première condition : le climat vraiment que les élections locales sont aujourd'hui la première préoccupation de nos concitoyens et que le renouvellement des présidents des conseils régionaux et départementaux soit leur priorité ? On peut en douter. Selon moi, ils aspirent davantage à sortir de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, ainsi qu'à retrouver leur vie d'avant.

Pensez-vous que tout le monde a accès à une campagne numérique, surtout en milieu rural ? Que tous les candidats aux départementales auront droit à un débat télévisé ? Non Certains doutent d'une réelle légitimité des personnes élues si l'expression du pluralisme n'a pu avoir lieu, si l'accès à la notoriété n'a pas été égal. Troisième condition : l'organisation du scrutin, ainsi que les modalités concrètes permettant de le mettre en place. Bien sûr, vous avez raison, la France ne peut être le seul pays à ne pas pouvoir voter. Mais le conseil scientifique a indiqué que, si les élections devaient se dérouler, un protocole renforcé serait nécessaire, avec les contraintes que nous connaissons : celles-ci devront être portées à la connaissance de ceux qui seront chargés d'organiser les opérations de vote, c'est-à-dire les maires. C'est pourquoi je salue la consultation des maires de France, auxquels nous allons demander d'assumer l'organisation

Je le regrette, car elle a été organisée à la suite des nombreuses craintes exprimées par les territoires. Sans aucune intervention de ma part, le département dont je suis l'élu a d'ailleurs majoritairement voté pour un report

Le taux de réponse massif a bien montré que l'unanimité n'était pas celle qui a été avancée par les instances représentatives. La réponse des maires est l'expression de craintes justifiées et d'exigences auxquelles il nous faudra répondre. Leurs propositions, d'ailleurs pertinentes, seront entendues et prises en compte. J'entends bien

D'autres pays ont voté dans des conditions variées, avec des taux de participation très différenciés. J'entends que la démocratie doit être respectée. Tous ces arguments sont fondés. Si nous sommes en mesure de répondre à l'ensemble des interrogations, si un consensus se dessine avec les associations représentatives, les partis et les mouvements, le Gouvernement reprendra les propositions dans la loi qui sera votée. Le scrutin peut être envisagé en juin. Nous y sommes

le Gouvernement devra prendre toutes les mesures, certaines déjà évoquées et d'autres à venir. Je pense à la transmission aux maires d'un guide régulièrement mis à jour relatif à l'organisation du scrutin la mise à la disposition des candidats d'un kit de campagne numérique ; ou, le jour du scrutin, à la mise en place de plages horaires préférentielles pour les publics vulnérables, les personnes contaminées ou susceptibles de l'être. Ces mesures permettront une campagne digne,

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, les juristes aiment user de locutions latines pour caractériser telle ou telle règle de droit ou situation atypique,

Nous sommes légitimement en droit de nous interroger sur l'intérêt d'utiliser, une fois de plus, l'article 50-1 de la Constitution, que nous avons encore eu l'occasion d'apprécier il y a quelques jours. Pour tout vous dire, nous autres parlementaires ne savons plus s'il faut considérer que nous sommes là pour entériner symboliquement des décisions déjà prises dans des enceintes plus confidentielles, ou si nous servons d'excipient pour mieux diluer la responsabilité de décisions que l'exécutif ne souhaite pas nécessairement endosser dans sa globalité. Bien sûr, personne ne niera la difficulté de votre tâche, monsieur le Premier ministre, ni même la complexité de décider sous la pression d'une opinion publique fatiguée et d'élus parfois versatiles, y compris parmi vos plus proches soutiens. Nous en avons bien conscience Pour autant, je vais vous répéter exactement ce que je vous disais il y a une semaine à cette tribune : nous n'avons pas la même définition du choix collectif dans une démocratie parlementaire. Or, au fond, ce dont nous débattons aujourd'hui n'est rien d'autre que la question fondamentale pour notre société de sa continuité démocratique dans des circonstances exceptionnelles. Nous avions déjà abordé cette question l'année dernière à l'occasion du report des élections municipales.

Dans notre conception d'une République moderne et transparente, nous aurions souhaité que toutes les options relatives au calendrier électoral soient mises d'emblée sur la table, nonobstant toutes les incertitudes liées à l'évolution de la situation pandémique, en particulier lors de nos débats sur la loi du 22 février dernier. Cela aurait sans doute évité les effets désagréables d'une consultation des maires précipitée en un week-end- quand bien même elle aura eu le mérite d'exister et de donner une voix à ceux qui se retrouveront une nouvelle fois en première ligne, pour organiser le scrutin dans les meilleures conditions possible. Je tiens d'ailleurs à saluer la grande réactivité des maires de France dans l'Hexagone et en outre-mer, qui ont été près de 24 000 à répondre à cette consultation, quel que fût le sens de leur réponse, en à peine quelques heures. Je n'oublie pas non plus l'implication des associations d'élus, dans toute la diversité de leur expression. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, puisque je vous en ai fait part par courrier la semaine dernière, mon groupe est avant tout viscéralement attaché au respect, en toutes circonstances, des principes fondamentaux de notre vie démocratique, qui doivent régir aussi bien la régularité du déroulement de la campagne électorale que la sincérité du scrutin et l'égalité entre tous les candidats. Or, vous en conviendrez, il n'existe pas à ce jour de solution idéale à même de garantir un déroulement normal du scrutin, que ce soit juridiquement ou politiquement, dès lors que les conditions sanitaires qui seront celles du mois de juin prochain sont incertaines. Faut-il alors lâcher la proie pour l'ombre ? Nous ne le pensons pas, et je vous confirme que mon groupe se ralliera dans sa majorité à l'idée de maintenir les deux scrutins en juin prochain.

L'urgence d'un retour à une vie normale se fait sentir partout. Nous y incluons évidemment l'urgence de la continuité démocratique, car si l'on peut maintenir les entreprises ouvertes, les bureaux de vote peuvent l'être aussi. Monsieur le Premier ministre, nous y attachons d'autant plus d'importance que le plus grand risque, nous le savons tous, est celui d'une abstention massive de nos concitoyens. Cette abstention serait encore plus significative

pour que l'abstention ne soit pas le premier parti de France, ouvrant la voie à une légitimation des extrémistes ! Dans ces circonstances, comme l'ont relevé de nombreux maires consultés, il convient de s'appuyer sur l'expérience du renouvellement des conseils municipaux l'année dernière. Nous disposons aujourd'hui d'élus et de personnels municipaux parfaitement formés et réactifs. Je n'imagine pas un électeur se rendre dans un bureau de vote sans utiliser du gel hydroalcoolique ou respecter les distances. Les gestes barrières font désormais partie de notre quotidien. Nous considérons, par conséquent, que les mesures que vous avez annoncées vont dans une direction satisfaisante, quand bien même elles n'apportent pas de garanties absolues : report d'une semaine du scrutin- il coïncidera avec le départ du Tour de France

Pour autant, je ne veux pas oublier les réticences des quelque 40 % de maires favorables à un report, qui attendent notamment qu'une plus grande partie de la population ait été vaccinée. Quoi qu'il en soit, il importe par-dessus tout que l'égalité entre tous les candidats soit garantie. À ce sujet, soyons clairs : l'interdiction de toutes les réunions en intérieur comme en extérieur donnera à cette campagne électorale une nature singulière, comme un air de démocratie en quarantaine. De même, la centralisation des professions de foi sur un site internet soulève encore une fois la question de l'égal accès de nos concitoyens à cette information indispensable pour éclairer leur choix. Nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure, lors de la discussion de la proposition de loi du RDSE relative à la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique. Mes chers collègues, j'attire encore votre attention sur les conditions particulières dans lesquelles se dérouleront les scrutins dans les petites communes rurales,

Il conviendra de réfléchir à des solutions opérationnelles, avec le soutien de l'État. Monsieur le Premier ministre, c'est avec la conviction profonde que nous devons approfondir sans relâche ce qui nous relie tous,

à juin 2021 des élections des conseils départementaux et régionaux. Aussi, nous pouvons être surpris de l'organisation de ce débat suivi d'un vote au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Le développement économique, l'aménagement du territoire, les collèges, les lycées, les solidarités sociales et territoriales : autant de compétences exercées par les conseils régionaux et les conseils départementaux qui font au quotidien la vie des Françaises et des Français. Oui, monsieur le Premier ministre, la vie démocratique est exigeante. Elle est de la responsabilité de chacune et de chacun. Personne ne peut se défausser de sa responsabilité quant à sa mise en oeuvre.

Nous sommes donc réunis une nouvelle fois pour débattre de la tenue des élections départementales et régionales. Personne ne découvre qu'il y aura cette année deux scrutins à organiser le même jour. Nous le savons depuis la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.

de partir des réalités du terrain, pour prendre les meilleures décisions et garantir que, partout sur le territoire de la République, les campagnes électorales et les élections puissent se tenir. dès la promulgation de la loi du 22 février dernier, vous pouviez organiser une consultation des maires sur les modalités du report et l'organisation du scrutin, un scrutin qui, je le rappelle, rassemble deux élections le même jour. le même jour. Les groupes parlementaires et les formations politiques auraient apprécié d'avoir ce retour du terrain, fruit d'un travail de concertation de plusieurs semaines, avant de vous remettre nos contributions le 8 avril dernier. De fait, monsieur le Premier ministre, le référendum express du week-end dernier ne peut être assimilé à une consultation. Mais nous nous souviendrons de votre capacité à pouvoir informer et consulter en un temps record l'ensemble des maires de notre pays ... Ainsi, les difficultés rencontrées ces derniers mois dans la relation avec les élus locaux, souvent mis devant le fait accompli, ne se reproduiront plus ! Nous sommes donc rassurés quant à la capacité de votre gouvernement à consulter les élus locaux,

de ce débat, nous voulons rappeler qu'une élection démocratique se déroule en trois moments importants : la campagne, le vote et le dépouillement.

tous les candidats en ont pris acte. Ce temps de rencontre avec nos concitoyennes et concitoyens, de confrontation des idées et d'incarnation des propositions par les candidates et les candidats demeure indispensable.

Demeure toutefois la question des élections départementales, qui sont tout aussi importantes que les élections régionales. C'est vrai ! Là encore, les médias, dans leur diversité, doivent rendre visibles non seulement les compétences du département, mais encore le débat démocratique au sein de chaque canton. le vote, nous savons d'ores et déjà que les maires ont à coeur que toute la sécurité soit assurée. Il faut donc travailler jusqu'à la tenue du scrutin pour adapter les opérations de vote.

peut participer aux opérations de dépouillement, car nous avons de plus en plus de difficultés, dans nombre de communes, à trouver des scrutateurs. Il faudra également trouver des lieux suffisamment aérés et spacieux pour permettre la présence de plusieurs tables de dépouillement, afin de garantir la sincérité

Vous avez attendu le week-end dernier pour demander l'avis des maires. Vous nous annoncez aujourd'hui la mise en place d'un comité pluraliste visant à travailler sur les modalités d'organisation et la préparation d'un nouveau projet de loi pour permettre certaines adaptations, certes indispensables. Que de temps perdu pour arriver à une telle précipitation qui, oui, pourrait laisser penser que votre objectif initial n'était pas de tout mettre en oeuvre pour la tenue, en juin prochain, de ces deux scrutins Nous prenons acte de vos propositions ; nous vous rappelons votre responsabilité à l'égard de la santé des Françaises et des Français et du maintien de la démocratie locale. Vous nous demandez

parce que nous ne jouons pas avec les scrutins de façon politicienne, parce que nous avons le souci de la démocratie locale, qui ne doit jamais être confinée, nous voterons très majoritairement en faveur du maintien de ces deux scrutins, en vous demandant solennellement, monsieur le Premier ministre, de tout mettre en oeuvre pour en assurer la réussite démocratique.

Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté attentivement et je vous ai senti soulagé : soulagé que le calendrier adopté par le Parlement en février dernier soit respecté

sommes pour la démocratie française. Voyez-vous, j'ai la faiblesse de penser que la consultation des maires a été organisée avec le secret espoir que l'idée du report serait majoritaire. la faiblesse de penser que cette consultation a été organisée pour contourner l'avis de la majorité des corps intermédiaires- partis, associations d'élus, etc. -qui étaient favorables au maintien.

avec cette consultation, « caramba, c'est encore raté ! » Oui, nous sommes soulagés pour la santé de la démocratie française. Aujourd'hui, il s'agit non pas d'exprimer un point de vue d'opportunité, mais de prendre nos responsabilités. La grandeur de la politique, c'est d'exprimer des choses fortes et graves, indépendamment des intérêts du moment, des sondages et des aléas.

Monsieur le Premier ministre, je pense que c'est une nécessité ; c'est l'enjeu même de ces futures échéances électorales. Certes, en mars de l'année dernière, il pouvait être naturel de reporter le second tour des élections municipales, car nous n'avions que peu d'informations sur le virus, mais la chanson n'est plus la même aujourd'hui. Depuis plus d'un an, nous vivons quotidiennement avec le virus, les gestes barrières, les masques et les restrictions de liberté. Oui, notre vie est affectée par le virus, mais elle ne s'arrête pas et elle ne saurait être confinée. Il en va de même pour la démocratie : celle-ci ne peut pas s'arrêter. Je parlais, en introduction, d'une démocratie en bonne santé ; une démocratie en bonne santé, c'est le meilleur vaccin contre le populisme, contre l'extrémisme, contre les « passions tristes », comme le disait Spinoza. je crains qu'il nous faille plusieurs doses de ce vaccin ... Une démocratie en bonne santé, c'est tout d'abord le respect de nos institutions. Il faut que le Gouvernement écoute les parlementaires et les élus locaux.

pas ou plus à la décision, on les informe après coup, quand tout est fait. Quand j'entends le président du groupe Union Centriste, Hervé Marseille, dire, avec son sens de l'humour, que le meilleur outil du parlementaire est son poste de télévision, je souris, mais je m'inquiète aussi Nous avons tenté de vous tendre la main, de participer à la décision, mais notre démocratie est malade de ne reposer que sur un homme seul. C'est d'ailleurs le mal endémique de la V République, dans sa version « quinquennat Dans une démocratie en bonne santé, le citoyen ne peut pas se limiter à choisir son président, fût-ce Jupiter, une fois tous les cinq ans. Nos institutions, ce sont d'abord nos maires, les fantassins de la République,

de respect. Une démocratie en bonne santé, c'est également le respect des corps intermédiaires, des syndicats, mais aussi des associations professionnelles ou d'élus.

si leur réponse ne vous convient pas ou si vous n'avez pas confiance. Oui, les élus de la République sont politiques et font, par nature, de la politique, mais, non, cela ne veut pas dire que leur avis est intéressé ou ne mérite pas d'être entendu, surtout quand il a été sollicité. Je suis moi-même élu départemental de Dominique Bussereau, président de l'ADF, je vois que c'est quelqu'un qui est capable d'objectivité, apte à dire quand les choses vont dans le bon sens et à saluer les bonnes décisions, mais aussi à alerter, quand une décision pose problème ou est inacceptable. Les corps intermédiaires font partie des acteurs majeurs de notre démocratie et leur voix mérite d'être entendue et respectée. Une démocratie en bonne santé, c'est, enfin, une démocratie qui respecte les libertés fondamentales.

Il serait donc inconcevable qu'une grande démocratie comme la France ne soit pas capable d'organiser des scrutins électoraux. Voyez nos voisins européens, qui continuent de voter ! Voyez nos alliés historiques, de l'autre côté de l'Atlantique, qui organisent une élection présidentielle au plus fort de la pandémie ! Je ne peux pas imaginer que nous ne soyons pas capables d'organiser un scrutin territorial chez nous Évidemment, des mesures exceptionnelles sont à prendre, mais rien ne doit pouvoir arrêter le train de la démocratie. Penser que nous pourrions, pendant encore plusieurs mois, arrêter ce train reviendrait à sortir du cadre démocratique. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous êtes, de longue date, favorable au maintien de ces échéances et je vous en remercie. Votre rôle est aussi de veiller au respect des institutions et des principes qui régissent notre République. Lors d'un voyage personnel au Vietnam, j'avais été étonné par la réponse d'un guide à qui je demandais ce que cela lui faisait de vivre dans un régime militaire. Il m'avait répondu : « C'est simple,

c'est que la démocratie est en danger ! La démocratie, c'est beaucoup plus. C'est faire face ensemble, malgré les difficultés. Dans cette période trouble, la démocratie doit démontrer sa force, sa plus-value, son supplément d'âme. Elle ne peut pas montrer sa supériorité seulement par beau temps. Il doit aussi y avoir une démocratie par gros temps, une démocratie qui démontre qu'elle est le meilleur régime dans une tempête.

Les maires souhaitent que l'État leur donne des autotests et que des règles claires, mais non contraignantes, soient fixées pour les assesseurs et le dépouillement- vous en avez parlé dans votre intervention, monsieur le Premier ministre. Notre groupe votera majoritairement pour la tenue des élections en juin prochain, parce qu'il est lassé de ces débats permanents sur la modification des modes de scrutin, sur d'éventuels redécoupages ou encore sur des variations de calendrier. Pour améliorer sa santé, notre démocratie a besoin de calme, de stabilité, j'allais dire de sagesse. La grandeur de la démocratie, la légitimité des élus, c'est l'onction du suffrage universel, ce sont ces beaux dimanches de printemps, pendant lesquels les candidats montent sur la balance,

y a-t-il une stratégie gouvernementale en matière d'élection depuis un an ? En général, on préjuge que les décisions politiques reflètent une volonté, mais il existe, en sociologie, un autre modèle explicatif : celui de l'anarchie organisée, dans lequel les décisions sont le produit d'une combinaison aléatoire, et non d'un processus rationnel.

dernier épisode en date, celui de, avec une séance de poker menteur autour du maintien des élections en juin, tandis que des arrêtés préfectoraux pour le scrutin départemental étaient signés et des mémentos édités.

J'entends la difficulté des sujets à traiter pendant une période aussi particulière que celle que nous traversons depuis plus d'un an, ... J'en doute ... ... mais de deux choses l'une : soit les élections constituent un sujet véniel, soit, au contraire, elles sont un sujet substantiel. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a toujours considéré que la seconde position s'imposait et que, pour cette raison, il fallait anticiper, de la même manière qu'il faut anticiper d'autres scrutins. Comme le Président de la République l'a déclaré le 13 avril 2020- 2020, non de 2021 -, « cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ». Les démocraties sont des systèmes marqués par le choix populaire. On mesure mal la radicalité, à l'époque, du discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln, quand celui-ci déclarait que la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Ce faisant, il posait ce dernier comme unique source et arbitre du pouvoir. Si les citoyens ne sont pas placés en arbitre de toutes les compétitions électorales, alors c'est le système en tant que tel qui est remis en question. Reporter des élections, c'est suspendre l'essence de la vie démocratique. Or, si la démocratie ne se réduit pas au vote, il n'y a pas de démocratie sans vote. Les élections sont à la fois le tissu qui fait exister notre régime et la fabrique de celui-ci. Or, pour vous, le sujet électoral est devenu périphérique. Si tout le monde s'entend sur la primauté absolue des questions sanitaires, économiques et sociales dans la période actuelle, cela ne signifie pas pour autant que la vie démocratique doive disparaître en fond de décor, quoi, lentement, les libertés s'étiolent et il se construit une servitude qui, à défaut d'être volontaire, est sanitaire ... Savez-vous, monsieur le Premier ministre, que les droits et les libertés publiques ont reculé dans le monde en 2020 ?

Votre gestion électorale est à l'image de votre gestion de crise : erratique. On aurait espéré qu'il n'en soit pas ainsi et que ce que l'on perdait en matière de libertés publiques, on le gagnerait en efficacité ; ce ne fut pas le cas. Je serais injuste, en ne reconnaissant pas la nécessité du soutien à l'activité, sans lequel, il est vrai, notre économie se serait effondrée, mais vous n'avez toujours pas pris la mesure des difficultés sociales, notamment celles des plus jeunes, et notre plan de relance est l'un des plus limités des pays occidentaux.

dans la mise en oeuvre de la campagne de vaccination, dans un contexte dégradé, parce qu'un homme seul, dans une opacité qui défie l'entendement, a décidé d'une trajectoire sanitaire à contre-courant des pays qui nous entourent.

Plus fondamentalement, votre attitude dit quelque chose de votre rapport au territoire. Je pense réellement que, pour cette majorité, ces élections sont accessoires, sinon encombrantes, un peu comme le sont les corps intermédiaires et le Parlement ... C'est pour cela que le grand feuilleton du report a été lancé : il visait initialement, dans une vaine et triste tentative, à se débarrasser du scrutin, en

Cela permet de faire diversion, afin de ne pas aborder d'autres sujets plus importants, comme la stratégie vaccinale ou la réouverture de notre pays à la mi-mai, tout en cultivant le procès en déconnexion des politiques qui osent s'attarder sur le scrutin électoral. À dire vrai, vous êtes enfermé dans une conception présidentialiste absolue de la V République : seule l'échéance présidentielle vous obsède, vous ou le Président de la République. On peut comprendre, de l'extérieur, votre volonté d'enjamber les élections locales. En effet, pour la première fois depuis 1958, ce gouvernement et sa majorité ne procèdent de rien : ils ne procèdent pas d'un parti et encore moins de convictions. Le Gouvernement ne procède que du Président de la République et, comme il lui doit tout, la seule échéance qui compte est celle qui le concerne. Les élections locales deviennent alors, au mieux, des péripéties aménageables, au pire, des élections de second ordre. C'est sans doute ce qui explique votre désinvolture dans la façon dont vous avez consulté les maires, le week-end dernier, alors que le casse-tête du calendrier était connu depuis plusieurs semaines.

Cette consultation tardive, au-delà du manque de transparence, comme, semble-t-il, pour les données sanitaires, était orientée. Le deuxième point est lié au précédent : sauf exception et alliance, vous n'existez pas dans les territoires, ou si peu.

Ce dernier report d'une semaine, comme une dernière boutade après tant de paris ratés, aura potentiellement de vraies conséquences en matière de participation, sous couvert d'un motif sanitaire. Cela constitue pourtant l'essentiel de vos aménagements, avec un comité de suivi. Le reste figure déjà dans la loi ou le règlement, voire est prévu de longue date- je pense notamment à la plateforme Ma Procuration. Vous nous annoncez de nouvelles mesures législatives à la marge- un dernier coup, sans doute, dans votre stratégie de brouillage.

Il n'est pas possible de dire aux Français qu'ils peuvent travailler et consommer, mais qu'ils ne peuvent pas voter, ce dernier geste prenant pourtant, en général, moins de temps. Il n'est pas possible de ne pas adapter les campagnes électorales et le vote de manière structurelle, alors que d'autres pays l'ont fait. Vous avez pourtant refusé de le faire. Avec constance, sur tous les textes ayant trait aux sujets électoraux, nous avons porté une multitude de propositions, comme nous le faisons sur d'autres aspects de la crise. Nous le faisons depuis un an au travers d'amendements, dont, par mansuétude, je tairai le nombre, et de propositions de loi,

Vous avez noyé la réflexion sur le vote par correspondance sous des considérations communautaires. Pourtant, le conseil scientifique le défend. Lorsque, pour la énième fois, j'ai avancé cette proposition, Mme la ministre Schiappa m'a doctement répondu que « ce n'est pas parce que cela se fait ailleurs que c'est forcément bien. tout de même avec les autres démocraties qui, autour de nous, ont su s'adapter avec efficacité et célérité ! Même le vote sur trois jours n'a pas trouvé grâce à vos yeux ni d'ailleurs à ceux de la droite sénatoriale. La mobilisation des médias audiovisuels pour la campagne a été rayée par votre majorité parlementaire avant que vous ne reveniez à de meilleurs sentiments. La campagne d'information que vous évoquez n'est autre qu'une proposition du Sénat qui, elle, au moins, aura été préservée. Nous vous avons même suggéré des bureaux de vote en extérieur, ce que la circulaire du 18 juin 2020 prévoit déjà. Dans tout cela, la diversion fonctionne, au détriment du fond et du débat démocratique qui s'abîme. Monsieur le Premier ministre,

c'est que, s'il n'était pas trop tard, beaucoup de choses auraient dû et auraient pu être préparées plus tôt pour concilier exigences démocratiques et sanitaires.

parole est à M. Jean Louis Masson, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

Malgré cela, le Gouvernement a essayé de passer outre, en organisant une pseudo-consultation des maires dans des conditions tout à fait scandaleuses. Afin d'empêcher un vrai débat sur le sujet, l'opération a été préparée dans le plus grand secret, sans que personne

compte tenu de la coupure du week-end, les maires étaient dans l'impossibilité d'avoir une vision contradictoire et de connaître les arrière-pensées de cette consultation faussement démocratique. En réalité, cette manoeuvre est digne d'une république bananière le Gouvernement espérait que, faute d'information et de débat, les maires se laisseraient faire, se laisseraient abuser. Heureusement, ceux-ci ont bien réagi une majorité claire, pour le respect de la démocratie, donc pour le maintien de la date des élections, à l'instar de ce qui a été fait dans tous les autres pays européens. Il s'agit d'un

Par ailleurs, lors des précédents débats parlementaires, j'avais demandé que, comme par le passé, ce soient les services préfectoraux qui se chargent de l'envoi des professions de foi et des bulletins de vote. Je regrette que la commission des lois du Sénat n'ait pas retenu mes amendements à ce sujet. En effet, compte tenu des délais, l'un des deux opérateurs retenus- la société Adrexo -craint d'avoir des difficultés pour acheminer correctement les professions de foi vers les électeurs. Cela confirmerait qu'il faut absolument revenir à l'ancien système, qui fonctionnait correctement. En tout état de cause, il y aura probablement de graves dysfonctionnements dans l'envoi des professions de foi en juin prochain et cela m'inquiète. C'est d'autant plus préoccupant que, compte tenu des restrictions liées à l'épidémie de covid, les professions de foi joueront dans la campagne électorale un rôle beaucoup plus important que ce que l'on a connu par le passé.

Chacun consultera ses agendas

également profiter de cette ultime intervention devant vous pour clarifier ce qui mérite encore de l'être. D'abord, je veux vous dire de la façon la plus claire possible que je partage avec vous- je sais que vous n'en doutez pas

De la même façon, mesdames, messieurs les sénateurs, nous respectons la démocratie, les maires et ce que vous avez appelé « les corps intermédiaires », notamment les associations d'élus.

des équilibres constitutionnels et des institutions de la V République que je respecte et dont j'ai toujours soutenu les principes, ce que je revendique devant vous.

À la demande du Gouvernement, le Sénat est appelé à se prononcer par un vote sur la déclaration

Plus personne ne demande à voter ? ... Le scrutin est clos.

résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du

Dans la discussion générale, la parole est à M. Éric Gold, auteur de la proposition de loi. Madame la Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, carte d'identité, permis de conduire, certificat d'immatriculation : pour ces titres, les procédures de délivrance sont désormais dématérialisées. Les usagers ne doivent plus se rendre en préfecture ; ces démarches administratives s'opèrent exclusivement en ligne. Cette modernisation répond aux attentes de nombreux usagers, qui accueillent favorablement la praticité, la célérité et l'efficacité des services publics. Mais l'évolution n'est pas reçue de la même manière par tous elle révèle en effet une inégalité face à l'usage des outils numériques, puisque 14 millions de Français ne les maîtrisent pas. Cet illectronisme touche particulièrement les populations les plus fragiles les personnes en situation de handicap, les personnes illettrées, les personnes détenues, les personnes sans abri ou encore les étrangers, comme l'a souligné le rapport d'information de notre ancien collègue Raymond Vall- je tiens d'ailleurs à saluer le travail qu'il a réalisé dans le cadre de la mission d'information présidée par Jean-Marie Mizzon. Outre l'exclusion par la compétence demeure l'exclusion matérielle, qu'elle soit due à une couverture numérique insuffisante ou à un manque d'équipement. En matière de connexion internet, seulement 50 % de la population ultramarine est raccordée et le nombre de maisons de services au public est insuffisant par rapport aux besoins. La fracture numérique existe encore et se superpose à la fracture territoriale, créant des « déserts administratifs ». Les territoires situés en zone blanche sont le plus souvent ceux qui ont subi auparavant la disparation de leurs services publics de proximité et le désengagement de l'État. L'objectif visant à dématérialiser l'ensemble des 250 démarches administratives les plus utilisées d'ici à 2022 soulève des inquiétudes légitimes au sein de la population et des élus. Le Défenseur des droits avait démontré dans son rapport de 2019 un recul de l'accès aux services publics et donc de l'accès aux droits. Cela n'a rien de surprenant, lorsque l'on sait que, d'après l'Insee, 60 % de la population serait incapable de réaliser des démarches administratives en ligne. Ce phénomène risque de s'accroître si rien n'est fait pour permettre l'inclusion numérique de tous nos concitoyens sans exception. La modernisation de l'État par la dématérialisation des services publics est une conséquence du principe d'adaptabilité et de mutabilité du service public. Celui-ci implique de réaliser des efforts considérables en matière de formation au numérique à tous les niveaux, par l'école et les entreprises. Ce principe exige une médiation numérique afin de favoriser l'autonomisation de l'usager ou, lorsque cela s'avère nécessaire, son accompagnement. Les initiatives sont nombreuses, mais elles n'ont pas encore permis d'atteindre les objectifs fixés. Les pass numériques devant servir à financer la formation numérique sont déployés à un rythme trop lent et ont une valeur insuffisante. L'organisation des lieux de formation au numérique souffre d'un manque de lisibilité, si bien que l'on assiste aujourd'hui à un empilement de structures développées de manière non coordonnée. Le principe d'égalité devant le service public commande de garantir l'accès de tous nos concitoyens à un accueil physique et de préserver la possibilité de ne pas recourir à des démarches dématérialisées lors des échanges avec l'administration. Certaines situations complexes nécessiteront une intervention humaine et un maillage fin des services publics sur l'ensemble du territoire. Afin d'offrir une solution aux 14 millions de Français qui souffrent d'illectronisme et d'atteindre l'objectif d'une inclusion numérique pour tous, j'ai déposé, avec plusieurs de mes collègues du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, cette proposition de loi qui entend traduire une partie des préconisations de la mission d'information du Sénat. Parce qu'il est fondamental de disposer d'un état des lieux précis de l'illectronisme pour guider l'action publique, le chapitre I de la proposition de loi prévoit deux mesures. L'article 1, prolongeant l'initiative conduite par l'Insee, propose de procéder à une évaluation biannuelle des capacités numériques de nos concitoyens à partir d'un référentiel commun. Afin de détecter en amont les publics fragiles, l'article 2 introduit la réalisation d'un test d'évaluation des compétences numériques lors de la Journée défense et citoyenneté. Les évaluations existent déjà, mais elles ne reposent pas sur un référentiel commun unique permettant de suivre l'évolution de la maîtrise des compétences numériques dans le temps. Le chapitre II a pour objectif de rendre les services publics 100 % accessibles,

Je tiens à préciser que nous sommes favorables à cette dématérialisation. Nul ne saurait revendiquer le retour au papier, mais les supports traditionnels doivent venir en complémentarité. Les maisons France Services peuvent répondre aux attentes de certains de nos concitoyens, mais ne peuvent pas toujours apporter une solution pour des dossiers de fond. Dans cette perspective, l'article 3 précise que tout usager doit bénéficier d'un « droit au guichet pour la réalisation de toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard dans les deux mois à compter de la date de la saisine. Cet article reprend une proposition du Défenseur des droits. L'article 4 prévoit une liberté de choix de l'usager des services publics en ce qui concerne les moyens de correspondance et de paiement. En outre, les décisions les plus importantes, celles d'attribution ou de révision des droits comportant des délais et des voies de recours, devront être notifiées sur support papier ou électronique selon le choix de l'usager. L'article 5 reconnaît un droit à l'erreur lors de la réalisation d'une démarche dématérialisée en cas d'erreur de saisie. L'article 6 dispose que l'accès aux sites internet des administrations et les téléservices doivent gagner en ergonomie. Cela vise à garantir la parfaite information des usagers et à faciliter l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs. Il est donc proposé de créer un référentiel d'ergonomie garantissant notamment la possibilité de rectifier à tout moment les dossiers en cours avant leur dépôt, la délivrance d'un accusé de connexion et la possibilité de contacter le service compétent en cas de difficulté. Les sites internet doivent également être rendus accessibles aux personnes en situation de handicap : c'est l'objet de l'article 7. Le retard en la matière étant inacceptable, les sanctions sont renforcées en vue d'accélérer la mise en conformité des sites, qui était prévue pour 2012. En outre, le recours à la dérogation pour « charge disproportionnée » sera limité aux petites collectivités locales. Le chapitre III est consacré au financement de la politique d'inclusion numérique. L'article 8 instaure un fonds de lutte contre l'exclusion numérique, doté d'au moins 500 millions d'euros par an, ainsi qu'un chèque-équipement, sous condition de formation, à destination des ménages modestes. Les 250 millions d'euros prévus par le Gouvernement pour l'inclusion numérique dans le cadre du plan de relance, bien qu'inédits, sont insuffisants au regard du milliard d'euros recommandé par la mission d'information. L'article 9 prévoit que ce fonds sera essentiellement alimenté par les recettes de la taxe sur les services numériques dite taxe GAFA, ainsi que par le budget général de l'État. Il permettra le financement du pass numérique et le renforcement de son montant, la formation au numérique sur l'ensemble du territoire, la structuration d'une offre de médiation numérique de qualité, la couverture intégrale du territoire en lieux d'accompagnement numérique des usagers du service public, ainsi que le financement du chèque-équipement nouvellement créé. Le chapitre IV est relatif à l'accompagnement des usagers exclus de la dématérialisation des services publics. L'article 10 confie à l'Agence nationale de la cohésion des territoires la charge d'établir une cartographie de l'ensemble des lieux d'accompagnement des usagers et de guider la structuration de l'offre de médiation numérique sous un label unique. Il complète ainsi la stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée à la loi du 10 août 2018 L'article 11 dispose que les établissements publics de coopération intercommunale désignent un référent « inclusion numérique » chargé d'accompagner et de coordonner les initiatives locales en matière de médiation numérique. Ce référent constituera un point de contact pour le secteur associatif. Le chapitre V comporte des mesures visant à renforcer la formation des élèves, des enseignants, des salariés et des dirigeants des entreprises. L'article 12 consacre l'illectronisme, à l'instar de l'illettrisme et de l'innumérisme, comme priorité nationale prise en compte par le service public de l'éducation et les personnes assurant une mission de formation ou d'action sociale.

L'article 14 propose un crédit d'impôt au bénéfice des PME afin de permettre la déduction de 50 % des dépenses de formation au numérique de leurs dirigeants et salariés. Au sein des 120 millions d'euros accordés par le Gouvernement à ces entreprises, nous aimerions connaître la pondération des sommes destinées à la formation au numérique. Nous craignons en effet que la transformation numérique des entreprises et le développement de la vente en ligne n'absorbent l'essentiel de l'enveloppe. L'article 15 propose une entrée en vigueur de ces dispositions dans les six mois suivant la publication de la loi. Enfin, l'article 16 constitue le gage de la proposition de loi.

à la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique déposée par notre collègue Éric Gold et inscrite à l'ordre du jour de l'espace réservé du groupe RDSE. Elle fait suite au rapport du 17 septembre 2020 de la mission d'information du Sénat sur la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique et a pour objet d'offrir une traduction législative aux propositions En premier lieu, je tiens à indiquer que les travaux que j'ai conduits ont très largement corroboré l'actualité et la pertinence du constat opéré par le rapport de la mission d'information : l'ancrage profond du numérique dépasse le simple défi technologique pour poser, aujourd'hui, de profonds problèmes de société. Comme l'indique le rapport, « 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique et près d'un Français sur deux n'est pas à l'aise. Si la France est dans la moyenne européenne, la situation n'est pas satisfaisante. Les personnes en situation de handicap, qui représentent une personne en exclusion numérique sur cinq, subissent une double peine. Si les sites en ligne doivent être théoriquement accessibles, seulement 13 % de démarches administratives leur étaient,

a formulé une série de quarante-cinq propositions réparties en sept axes afin de lutter contre ce phénomène sous tous ses aspects. Ces axes comportent notamment l'évaluation de l'exclusion numérique, le passage à une logique « 100 % accessible » ou la construction d'une « éducation nationale 2.0 ». De son côté, le Gouvernement a mis en oeuvre plusieurs mesures de soutien financier pour favoriser l'inclusion numérique, notamment à travers le plan de relance instauré pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire actuelle. Ainsi, 120 millions d'euros sont consacrés dans ce plan à la numérisation des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises Par ailleurs, pour garantir un accès physique des usagers aux administrations, le Gouvernement a également créé un réseau de maisons labellisées « France Services », lesquelles vont progressivement remplacer les maisons de services au public créées en 2015. Ces structures sont des guichets uniques permettant aux citoyens de réaliser des démarches administratives relevant par exemple du ministère de l'intérieur, de la Caisse nationale des allocations familiales ou de l'assurance maladie. Elles assurent également un accompagnement numérique pour la réalisation des démarches en ligne. Au 1 février 2021, on comptait 1 123 maisons France Services

En outre, le Gouvernement a développé la plateforme Aidants Connect qui facilite l'intervention d'un tiers pour accomplir des démarches en ligne pour le compte d'une personne en difficulté. Afin de mettre en oeuvre les propositions du rapport d'information précité, la présente proposition de loi comporte seize articles répartis en quatre chapitres, que vient de vous présenter son auteur principal. Comme vous le savez, j'ai proposé à la commission des lois de ne pas adopter le texte au stade de la commission et je remercie celle-ci de m'avoir suivi.

de vous présenter, aujourd'hui, dans son espace réservé, une proposition de loi conforme à ses attentes, sur un sujet qui lui tient à coeur. En effet, à l'issue des travaux que j'ai conduits, je ne pense pas que la commission des lois pouvait adopter un texte sans modifier profondément la proposition de loi dont elle était saisie. plusieurs dispositifs ne relèvent pas de la loi ordinaire ou ne justifient pas une inscription dans la loi au regard de l'article 34 de la Constitution. D'autres soulèvent de vraies questions, mais n'offrent pas de véritables garanties. En tant que législateurs, nous sommes les premiers à savoir que les « coups de baguette législative » n'existent pas et qu'il est parfois plus efficace d'y substituer notre pouvoir de contrôle. Comme je l'avais indiqué au stade de la commission, je vais aujourd'hui vous présenter des amendements dont le but est de sécuriser cette proposition de loi en tant qu'instrument de droit. L'ampleur des suppressions suppressions et modifications que je vais vous proposer ne doit pas trahir la volonté de la commission des lois. Certes, ces amendements pointent des faiblesses juridiques, mais ils n'occultent pas l'occasion qui est aujourd'hui donnée de débattre d'un sujet majeur. Cet examen permettra, d'une part, de faire un point sur les conclusions de la mission d'information qui a rendu ses travaux il y a quelques mois. d'autre part, l'opportunité d'entendre le Gouvernement nous présenter, au fil des débats, l'ensemble des mesures qu'il a mises en oeuvre pour lutter contre l'illectronisme, notamment en cette période d'isolement et de crise sanitaire. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir chaleureusement remercié Éric Gold et nos collègues du groupe RDSE, qui nous permettent

numérique. Nos débats seront l'occasion de rappeler l'action continue et approfondie du Gouvernement en faveur de cette politique. Je tiens également à saluer très sincèrement le travail de fond que les sénateurs ont mené, contribuant directement à donner de la visibilité à une réalité trop souvent oubliée, celle de l'illectronisme. Nul besoin de rappeler, de rappeler, vous le savez aussi bien que moi, la place croissante que prend le numérique dans nos vies de citoyens, de consommateurs, de travailleurs, de parents, d'étudiants. Cette révolution numérique bouleverse fortement le quotidien des Français. Elle implique autant de risques

d'offrir les moyens de s'y acclimater. Nous connaissons tous dans nos entourages des personnes qui ont appris au gré de leurs motivations personnelles : les grands-parents pour maintenir le lien avec leurs petits-enfants ; les télétravailleurs confrontés aux outils de visioconférence ; les artisans et les commerçants, qui se sont

Face à ce constat, nous agissons concrètement et résolument depuis 2017, d'abord sur la qualité de la dématérialisation. Permettre aux Français de réaliser leurs démarches administratives du quotidien en ligne

et nous devons faire mieux. Pour cela, nous mobilisons des moyens inédits : 500 millions d'euros du plan de relance sont dédiés à la numérisation des administrations.

fonde sur une stratégie partenariale et collective- vous en rappelez l'importance dès l'article 1 de la proposition de loi -, coconstruite avec les collectivités territoriales, les opérateurs de service public, les acteurs de la médiation numérique et du travail social, ainsi que les entreprises. Le plan France Relance a accéléré de manière inédite cette dynamique. Aujourd'hui, 250 millions d'euros sont mobilisés pour les maisons France Services. L'objectif- nous venons de l'évoquer -est de mieux accompagner les Français dans leur quotidien.

Il s'agit d'abord d'encourager les collectivités locales à mettre en place des solutions numériques collectives, comme les plateformes de commerce local, dont nous avons pu mesurer l'importance depuis un an à l'occasion de la pandémie. Il s'agit aussi de s'adresser directement aux TPE qui souhaitent entamer une transformation numérique ; du chèque numérique de 500 euros proposé à toutes les entreprises de moins de onze salariés. Enfin, il va de soi que la lutte contre l'illectronisme passe par l'éducation

que l'expérience du premier confinement ne nous ait pas permis d'éviter les nombreux dysfonctionnements observés lors de la reprise de l'école à distance mardi dernier. Si nous avons eu la preuve durant cette période que l'outil numérique pouvait être une alternative aux rencontres en présentiel,

France urbaine et périurbaine, proche des centres de décisions, des services publics et des pôles économiques ; d'autre part, une France rurale, éloignée de tout, mais souvent plus conforme à la réalité de notre pays. Plus que d'égalité, c'est de justice et d'équité dont nous avons besoin pour renouer avec la promesse républicaine. À mon sens, cette proposition de loi y contribue.

Entre la maîtrise des réseaux sociaux et celle de l'outil informatique pour effectuer des démarches administratives, il n'y a qu'un pas, souvent trop grand pour de nombreux jeunes. À propos des articles 3 à 7 de la proposition de loi,

Elle doit également s'accompagner d'un droit à l'erreur, comme cela est proposé à l'article 5. Enfin, pour être acceptée, la dématérialisation doit être facilitée, notamment par une meilleure ergonomie des sites des administrations et une plus grande conformité aux normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Les dispositions proposées aux articles 6 et 7 nous permettent de faire un pas en ce sens. J'espère que nous trouverons un accord sur ces sujets. L'ensemble des membres du groupe du RDSE votera cette proposition de loi ; certes, elle ne résoudra pas tout, mais elle vient marquer une étape essentielle dans la lutte contre l'illectronisme. La

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous remercions vivement

Nous partageons totalement le constat global : « La dématérialisation de l'action publique ne doit pas aboutir à la suppression des guichets et à la déshumanisation du service public. Alors que le désir de vaccination occupe les esprits de tous nos concitoyens, nous mesurons, en tant qu'élus de terrain, les angoissantes difficultés qu'éprouvent certains d'entre eux pour obtenir un rendez-vous ou des informations sur les sites accessibles uniquement par les réseaux numériques. Nous sommes nombreux dans cette assemblée à leur avoir apporté un soutien essentiel pour leur permettre de profiter d'une aide qui aurait dû leur être fournie directement, sans l'intermédiaire d'un serveur informatique désespérément binaire. Combien de nos concitoyens âgés ne sont toujours pas vaccinés par défaut de connexion ou de maîtrise du numérique ? Bonne question ! D'une manière plus générale, nous remarquons, avec les auteurs de ce texte, que plus la dématérialisation des services progresse, plus elle abandonne à ses marges des populations qui se trouvent exclues par manque d'équipement, de compétence ou de réseau performant. Leur éviction de l'accès aux services publics numérisés les oblige souvent à recourir à des intermédiaires, qui leur font payer cette aide. C'est le retour de l'écrivain public qui vend ses compétences informatiques, comme jadis l'écrivain de rue faisait commerce de sa maîtrise de l'écrit et des formes d'interpellation des autorités publiques. De plus en plus, les collectivités apportent gratuitement ce service à leurs administrés menacés par l'exclusion numérique, y compris dans les territoires urbains, qui ne sont pas épargnés par un tel processus. Tout se passe comme si les administrations nationales reportaient sur les collectivités la charge de l'aide aux populations rejetées par une numérisation exclusive. Cette proposition de loi a le grand mérite d'alerter l'État sur les difficultés éprouvées par nos concitoyens et de rappeler justement l'importance du droit au guichet, tel que l'avait défini le Défenseur des droits dans son rapport de 2019. Néanmoins, elle ne peut pas contraindre l'État à mettre un terme à une dérive générale qui, par souci d'économie, remet en question la notion même de service public. Assurer une mission de service public, ce n'est pas délivrer une prestation technique dans l'ignorance volontaire des spécificités sociales ou territoriales des usagers. En déshumanisant de la sorte sa relation aux citoyens, l'État condamne le service public, parce qu'il le met en concurrence avec des services privés, qui n'ont pas les mêmes obligations de résultat. Une mission de service public se doit au contraire, au nom du pacte républicain, d'apporter une aide, une allocation, des droits adaptés à la situation personnelle de tous les citoyens, afin de n'en oublier aucun et de rendre effectif le contrat social qui nous unit au sein de la Nation. Nous voterons en faveur de ce texte dans l'espoir qu'il constitue la première étape d'une réflexion plus globale sur le rôle des services publics

parce qu'elle aggrave la situation des finances publiques sans prévoir de compensation équivalente. En outre, elle compte de nombreuses dispositions de nature réglementaire, comme l'a rappelé M. le rapporteur. Elle a cependant le mérite d'exister, et elle est particulièrement bienvenue tant il y a urgence à légiférer sur la fracture numérique qui frappe de plein fouet notre pays. Elle arrive dans le sillage du rapport du 17 septembre 2020 de la mission d'information du Sénat « Lutte contre l'illectronisme et inclusion numérique », que présidait notre collègue Jean-Marie Mizzon. Le constat y était accablant : 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique et près d'un Français sur deux n'est pas à l'aise avec cet outil de progrès Surtout, alors que la France compte 53 millions d'internautes, les plus âgés, les moins favorisés ou encore nombre de ruraux sont laissés pour compte dans une société toujours plus numérisée. Sans surprise, cette fracture sociale et générationnelle est aussi, dans une large mesure, territoriale. En effet, 50 % des non-internautes résident dans des communes de moins de 20 000 habitants. de mai 2018, la Cour des comptes avait évalué à 34 milliards d'euros le coût du plan France Très haut débit et estimé que l'objectif de raccordement d'ici à 2030 était nettement plus réaliste que la prévision initiale, c'est-à-dire 2022.

ligne. Pour toutes ces raisons, le passage d'une logique 100 % dématérialisée à une logique 100 % accessible semble, pour l'heure, quelque peu compromis. Fort de ces chiffres, le rapporteur de la mission, notre ancien collègue du Gers Raymond Vall, avait tenu à bien prendre la mesure de ce phénomène d'envergure, en précisant combien la lutte contre l'illectronisme dépasse largement le simple défaut de maîtrise technologique des outils numériques. De fait, l'illectronisme, qui peut aussi s'expliquer par un manque de compétences informatiques, provoque immanquablement une rupture d'égalité des citoyens,

C'est la raison pour laquelle le rapport demandait que l'inclusion numérique soit proclamée priorité nationale et service d'intérêt économique général.

Ne nous leurrons pas. L'argent est, ici plus d'ailleurs, le nerf de la guerre. Les propositions qui figurent dans le rapport, si elles sont mises en pratique, comme les actions menées jusqu'ici par le Gouvernement, donneront des des résultats uniquement si tout est mis en oeuvre au plan financier pour parvenir à un niveau d'inclusion numérique satisfaisant dans les meilleurs délais. À cet égard, égard, des préconisations du rapport, notamment de la proposition de professionnalisation de la médiation numérique ? Il y a pourtant là un vivier d'emplois qui pourraient séduire de jeunes diplômés, mais encore faudrait-il, là aussi, les rémunérer à leur juste valeur. Le SMIC, niveau ne peut décemment pas suffire. Dans ces conditions, puisque tout est une question de financement et de budget, de quels moyens le législateur dispose-t-il pour inciter le Gouvernement à agir au mieux et, surtout, au plus vite ? ? Et de cet ambitieux chantier d'inclusion numérique, décrété grande cause nationale ? Il est très attendu, en particulier dans nos territoires ruraux brusquement confrontés à la dématérialisation massive des services publics. La commission des lois a arrêté un périmètre indicatif pour cette proposition de loi. Celui-ci comprend la détection et l'étude des personnes en difficulté face au numérique, les échanges et procédures numériques avec l'administration, les compétences numériques (ANCT), la formation au numérique pour les personnels de l'enseignement et les aides en lien avec le numérique. Tâchons de nous y tenir, car il est un fait parfaitement établi et confirmé par la crise du covid-19 : la société numérique provoque l'exclusion de nombre de nos concitoyens.

les confinements ont jeté une lumière crue sur la détresse de 14 millions de personnes en situation d'illectronisme. Avec la digitalisation grandissante de notre société, les injustices sont exacerbées, et il y a une véritable rupture d'égalité. Pour beaucoup, travailler, étudier, accéder à ses droits et même se soigner devient un défi insurmontable. Car, outre que l'accès matériel au numérique est coûteux, son utilisation, loin d'être simple et intuitive, suppose d'en maîtriser les codes. Si dès 1999 Lionel Jospin pointait le risque d'illectronisme, encore aujourd'hui, près d'un Français sur deux n'est pas à l'aise avec le numérique, et près d'un sur cinq en reste totalement exclu. Ce qu'il faut appeler un échec est lié à l'absence de politique publique organisée. Notre conviction est qu'il faut envisager l'inclusion numérique comme un service public à part entière. Tout d'abord, ce service doit être structuré et organisé. Car, comme dans la lutte contre l'illettrisme, la difficulté de l'illectronisme réside dans la capacité à atteindre ceux qui en ont le plus besoin et qui nécessitent un accompagnement. Or les publics les plus éloignés du numérique ne sont ni repérés ni contactés. Parallèlement, l'atomisation des initiatives et la multiplication des niveaux décisionnels rendent les actions difficilement visibles pour les bénéficiaires. C'est pourquoi nous aurions souhaité qu'une telle compétence soit explicitement dévolue au département : compte tenu de sa mission de solidarité territoriale, de lutte contre les exclusions et d'accompagnement social, celui-ci apparaît comme l'échelon pertinent. Dans les faits, de nombreux départements se sont déjà saisis de cette problématique. Nous proposons ainsi que chaque département élabore un schéma de lutte contre l'illectronisme. Cela permettra de dresser un bilan des actions existantes sur le territoire, de mieux les coordonner et de les développer en fonction des besoins identifiés et en s'appuyant sur les structures existantes. Je pense notamment à La Poste, qui, grâce à son maillage territorial et à ses facteurs, couvre toutes les zones, même les plus reculées. Ainsi, la politique départementale de lutte contre l'illectronisme sera clairement définie, plus efficace et répartie équitablement sur le territoire. Ensuite, ce service public doit bénéficier d'un investissement à la hauteur de l'enjeu. Nous saluons à ce titre l'article 8, qui vise à instaurer un fonds de lutte contre l'exclusion numérique. De la même manière, l'article 9, qui permet aux ménages modestes de bénéficier d'un chèque-équipement pour l'acquisition de matériel informatique, nous paraît aller dans le bon sens. Cependant, il ne faut pas l'oublier : plus encore que le matériel, c'est le coût d'une connexion à internet qui est un frein. Il conviendrait de réfléchir à une aide pour le paiement d'un abonnement. Ces moyens doivent aussi permettre de développer la médiation numérique, encore insuffisante face à la dématérialisation des services publics. Si la liberté donnée à l'usager sur les moyens de correspondance et de paiement ou encore le droit à l'erreur sont bienvenus, c'est la question de la formation qui est primordiale, qu'il s'agisse des enseignants comme des élèves, des chefs d'entreprise comme des salariés. Nous soutenons donc les différentes mesures prévues dans le texte à cet égard. Afin que la formation puisse être efficiente, une bonne connaissance des besoins est essentielle. Nous considérons qu'une évaluation régulière des compétences numériques de nos concitoyens est loin d'être superfétatoire.

Enfin, le numérique ne doit pas être un facteur d'isolement pour les personnes en situation de handicap. Seuls 13 % des sites en lignes leur sont accessibles ; le renforcement des mesures pour accélérer la mise en conformité des sites semble nécessaire.

À ce titre, et parce que tout outil supplémentaire est utile pour lutter contre l'exclusion numérique, elle mérite d'être soutenue. La parole Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le vent de la révolution numérique est porteur de nombreuses promesses. Qu'il s'agisse du développement de l'accès à la connaissance, du renforcement de l'inclusion sociale ou de l'amélioration de la qualité de vie, voire de l'égalité territoriale, le numérique est à la croisée de tous les bouleversements. Pourtant, des inégalités flagrantes perdurent. Aujourd'hui, 14 millions de nos concitoyens sont confrontés à des difficultés dans l'utilisation des outils digitaux. Ce n'est pas rien ! Handicap, précarité économique, niveau d'instruction ... les causes de l'illectronisme sont multiples. Mais c'est à la problématique des seniors que je consacrerai l'essentiel de mon intervention. D'après les chiffres de l'Insee, près de la moitié des plus de 75 ans n'ont pas d'accès internet à leur domicile et 67 % d'entre eux sont dépourvus des compétences numériques élémentaires. Il n'est pas acceptable que nos aînés soient exclus de la marche du progrès. Il faut évidemment faire le nécessaire pour y remédier. Alors que le troisième confinement national et la généralisation de l'école en ligne nous ont fait franchir un nouveau palier dans la dématérialisation des relations avec l'administration, il est plus urgent que jamais de dessiner un cap pour garantir l'égal accès de tous les Français au service public. C'est la raison pour laquelle je soutiens le principe de la présente proposition de loi. Bien qu'émaillé de nombreuses imperfections juridiques mises en lumière par M. le rapporteur, ce texte a le mérite de proposer des solutions concrètes contre l'ostracisme numérique des populations les plus fragiles. Selon l'Observatoire des seniors, en 2014, 27 % des plus de 75 ans déclaraient souffrir de solitude. Il est primordial de veiller à ce que la dématérialisation n'accentue pas leur isolement. Et comment, par exemple, remplir sa déclaration d'impôts, lorsque l'on est isolé et que l'on ne dispose pas d'un ordinateur ? C'est pourquoi je salue la création des maisons France Services et de la plateforme Aidants Connect, qui facilite l'aide administrative de tiers aux personnes vulnérables. Plus largement, je voudrais en profiter pour souligner le travail remarquable accompli bénévolement par les aidants familiaux. Véritables anges gardiens du quotidien, des milliers de Français s'investissent sans compter au service de leurs proches les plus vulnérables.

Parler du grand âge, c'est aussi parler du handicap. Les personnes en situation d'invalidité représentent une personne sur cinq en exclusion numérique. Alors que les sites en ligne devraient théoriquement leur être accessibles, seulement 13 % des démarches administratives leur sont véritablement ouvertes sur internet. C'est pourquoi j'ai cosigné les amendements de Philippe Mouiller en faveur de l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. de handicap. Alors que nous vivons dans une société toujours plus dématérialisée, aucun citoyen ne devrait être sacrifié sur l'autel de la modernité. Le numérique pour tous est un enjeu d'égalité et même d'humanité ! La parole

collègues, cela a été rappelé, trois Français sur cinq rencontrent beaucoup de difficultés pour réaliser des démarches en ligne, 14 millions de Français sont éloignés du numérique et un Français sur deux déclare ne pas être à l'aise avec ces outils.

Loin d'apparaître comme un progrès, il peut être ressenti comme une entrave et conduire à des renoncements aux droits, ce que nous ne pouvons évidemment pas accepter. Il existe donc un véritable enjeu : s'adapter à la vie des Français, en prenant en compte leurs usages, qui passent effectivement de plus en plus par le numérique, mais pas de manière

De même, nous pouvons mentionner l'article 13, qui tend, d'une part, à rendre obligatoire la formation des enseignants des établissements d'enseignement supérieur en matière de numérique et, d'autre part, à prévoir que les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé) organisent la formation continue des enseignants en matière numérique. En effet, la définition du contenu matériel des enseignements que les Inspé dispensent relève plutôt du domaine réglementaire.

la nécessité de faciliter la vie de nos concitoyens sur le plan numérique. Toutefois, dans cette lutte contre l'illectronisme, les actions à mener ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi ordinaire

la secrétaire d'État, mes chers collègues, contraventions, impôts, sécurité sociale, puis, avec le confinement, télétravail, école à distance : le numérique s'est emparé avec succès, il faut le dire, de la relation du citoyen avec l'administration et, plus généralement, d'un grand nombre de domaines. Toutefois, si cette révolution numérique a eu un impact positif dans l'organisation de l'administration, les dysfonctionnements ne sont pas rares. À ce jour, chaque avancée du numérique s'accompagne encore d'un accroissement des disparités et des inégalités des citoyens face à ces outils et à leurs usages. tous vécu, je pense, des situations kafkaïennes, où, de réponse automatique en réponse automatique, plus aucun humain n'apparaît, aucun guichet n'est ouvert, aucun numéro de téléphone n'est à disposition pour que l'usager puisse résoudre ses problèmes administratifs. Ces dysfonctionnements touchent tout le monde, quel que soit le milieu social, économique ou culturel, mais encore plus les personnes détenues, les étrangers et les personnes illettrées. La précarité et l'âge creusent encore cette fracture. J'ai dit que nous étions tous concernés, mais ce « nous » englobe des situations bien diverses : manque de moyens financiers pour s'équiper ; coût des connexions à internet ; zones blanches ; absence de connaissances ou de formation ; difficultés de compréhension de ces outils. Tout comme l'illettrisme, c'est un fléau discret pour ceux qui en souffrent souvent de manière honteuse. Les personnes éloignées du numérique peinent en effet à demander de l'aide. La mission d'information du Sénat de septembre dernier avait pointé que « 14 millions de Français ne maîtrisaient pas le numérique » et que « près d'un Français sur deux n'était pas à l'aise ». Or la maîtrise de ces outils est devenue un paramètre incontournable pour l'accès effectif de l'usager non seulement au service public, mais aussi à l'emploi, voire, de plus en plus, à l'éducation, à la culture ou à l'information. La présente proposition de loi, que je salue, s'inspire de ce rapport et cherche, au travers de ses seize articles, à améliorer la situation actuelle, en permettant une meilleure prise en compte de ces publics en difficulté. le rapport sénatorial préconisait la mobilisation d'un milliard d'euros pour financer l'inclusion numérique, soit quatre fois plus que le montant alloué par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance. Je regrette que notre commission n'ait pas adopté ce texte, qui prévoit notamment un fondamental droit au guichet, essentiel dans la garantie réelle d'un accès au service public, un droit à l'erreur, notamment pour les aidants qui effectuent les démarches en ligne pour le compte de tiers, ou encore une compétence nouvelle pour l'Agence nationale de la cohésion des de médiation numérique sous une labellisation unique et établisse une cartographie de l'ensemble des lieux d'accompagnement des usagers du service public ». Enfin, dans son article 8, ce texte vise à créer un fonds de lutte contre l'exclusion numérique, doté d'au moins 500 millions d'euros par an, donc plus ambitieux que la stratégie nationale

Nous proposons également de permettre aux travailleurs sociaux, en première ligne dans la réduction de cette fracture, comme pour beaucoup d'autres sujets, d'être formés à la médiation numérique. Nous saluons et nous soutiendrons les démarches de nature à rappeler l'impact environnemental des outils du numérique et à garantir l'information de tous les nouveaux usagers sur cette

alors que nous vivons dans une société toujours plus numérisée, que nos démarches administratives tendent vers le 100 % dématérialisé, 14 millions de nos concitoyens éprouvent de grandes difficultés à se saisir des outils informatiques. L'illectronisme et les fractures numériques qui perdurent dans notre pays touchent un large public : les personnes âgées en premier lieu, mais aussi les personnes les moins diplômées, les ménages les plus modestes et même une partie de notre jeunesse, cette même jeunesse que l'on considère bien souvent comme étant à la pointe de la technologie, faisant fi de la diversité qui la caractérise. À l'heure où les offres d'emploi se trouvent majoritairement sur internet, où l'accès aux services publics et à l'information est dématérialisé, où le droit de saisine des administrations par voie électronique est devenu la norme, l'illectronisme éloigne nos concitoyens du monde du travail, freine leur émancipation et l'accès à leurs droits. Tendre vers une société numérisée est une ambition louable, partagée par les gouvernements successifs, mais, pour préserver notre pacte social et rendre le numérique accessible à tous, cette ambition implique des moyens. Des moyens en matière de formation : je pense notamment aux aidants, aux travailleurs sociaux, aux agents des collectivités territoriales et aux enseignants. Des moyens pour accompagner nos concitoyens les plus éloignés des outils numériques, afin qu'ils puissent s'en saisir pleinement et gagner en autonomie. Des moyens, enfin, pour permettre dans chaque territoire d'identifier les types de public en difficulté avec le numérique et de proposer l'offre d'accompagnement adaptée. C'est pourquoi, depuis 2018, l'État et les collectivités territoriales mettent en oeuvre la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Le plan de relance renforce cette stratégie ambitieuse : 250 millions d'euros seront ainsi mobilisés pour accélérer l'appropriation des nouveaux usages et services numériques par tous les Français. La proposition de loi que nous examinons s'inscrit pleinement dans la continuité du rapport d'information sénatorial rendu en septembre dernier ; nous en partageons le constat, ainsi que les objectifs. Ce texte contient des pistes d'amélioration intéressantes que je tiens à saluer. La reconnaissance à tout usager d'un droit à l'erreur lors de la réalisation d'une démarche administrative dématérialisée en cas d'erreur de saisie constitue une avancée notable, et l'élargissement de ce droit à l'erreur à un tiers agissant dans l'intérêt ou pour le compte de la personne en cause nous semble compléter utilement ce dispositif. Nous partageons également le constat sur la nécessité pour les sites internet des administrations de gagner en ergonomie. La création du référentiel, prévue à l'article 6, va dans le sens d'une meilleure information des usagers afin de faciliter l'exercice de leurs droits et devoirs. Il est aujourd'hui urgent d'accélérer la mise en conformité des sites internet pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap. Le retard pris en la matière compromet notre ambition commune de parvenir à une société inclusive et de favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi il est nécessaire de sanctionner les manquements aux règles relatives à l'accessibilité numérique, et non plus seulement l'absence de mention visible sur la page d'accueil. Enfin, la crise sanitaire a bouleversé nos modes d'enseignement et mis en lumière la nécessité de mieux former les enseignants aux outils numériques. L'article 13, qui prévoit la formation continue obligatoire des enseignants au numérique répond à cet objectif. s'agit de garantir une continuité pédagogique à tous les élèves et de leur offrir les ressources nécessaires pour appréhender les nouveaux outils numériques. Pour conclure, je tiens à saluer le travail de notre collègue Éric Gold, auteur de la proposition de loi, ainsi que celui de notre rapporteur, Thani Mohamed Soilihi, qui propose utilement de recentrer le texte sur les dispositions constituant un apport et ayant toute leur place dans une loi. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'inclusion numérique, ce sont des liens et des lieux. Liens humains d'abord, car c'est l'accompagnement par des médiateurs, des conseillers ou d'autres référents qui prime pour les 17 % de la population qui restent éloignés des usages du numérique et ne peuvent ni se relier au monde et aux administrations, de plus en plus distantes, ni accéder à leurs droits,

À ce propos, mes chers collègues, avez-vous déjà essayé de remplir vous-mêmes un quelconque formulaire administratif en ligne à l'aide d'un smartphone, qui plus est en zone blanche ? blanche ? Certains ont voulu nous faire croire, peut-être de bonne foi, qu'avec le suréquipement de nos concitoyens en téléphones dits intelligents la fracture numérique était en voie d'être réduite. La période que nous vivons actuellement nous prouve à quel point ils se trompaient. Parallèlement au déploiement des infrastructures télécoms fixes et mobiles- en même temps, si j'ose dire -, les collectivités ont accompagné les usages. Les élus locaux n'ont eu de cesse de mettre en place des lieux et de rémunérer des animateurs, que ce soient des cybercafés municipaux dans les années 1990, des points d'accès dans les mairies, les médiathèques ou les établissements scolaires ou encore des cyberbus. Certains de ces lieux et de ces postes d'animateur ont su s'adapter et survivre aux réorientations incessantes des politiques nationales. Nous pouvons donc nous réjouir aujourd'hui, plus de vingt ans après ces pionniers, qu'une stratégie nationale d'inclusion numérique soit de nouveau à l'ordre du jour. Nous ne pouvons que nous féliciter du fait que plusieurs centaines de millions d'euros lui soient enfin consacrées enfin consacrées et nous associer à cette grande cause nationale, notamment au travers de cette proposition de loi. Pour autant, plusieurs points de cette démarche sont perfectibles. Que pouvons-nous améliorer ? Premièrement, pour mieux détecter les publics en difficulté, il est essentiel de se mettre d'accord sur les données nécessaires pour définir un indice partagé entre État et collectivités, plutôt que d'adopter une classification stigmatisante, comme nous avons pu en entendre parler. Je me permets ici de faire référence au rapport sénatorial sur le devenir de La Poste, qui ouvre aussi certaines perspectives. Deuxièmement, il convient de passer du 100 % dématérialisé au 100 % accessible. L'ensemble des acteurs, dont les associations de collectivités, n'ont cessé de rappeler qu'il fallait, d'une part, laisser le choix à l'administré de son mode de relation avec l'administration et, d'autre part, offrir un mode d'accès alternatif, au mieux un guichet- les 2 000 maisons France Services annoncées vont dans ce sens -ou, pour le moins, un accès téléphonique avec des conseillers qui répondent. Troisièmement, le financement de la politique publique d'inclusion numérique devrait s'envisager sur le temps long. Il ne peut se satisfaire de incessants, voire contradictoires, au gré des changements gouvernementaux. Quatrièmement, sur l'accompagnement des usagers exclus de la dématérialisation des services publics, le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'ANCT, multiplie les actions et les appels à projets

Cette abondance de dispositifs permet d'aborder le problème de l'inclusion avec une palette d'outils, mais entraîne un inévitable problème de lisibilité, d'autant que, pour la plupart d'entre eux, le fonctionnement par appels à projets ne conduit bien souvent que les collectivités les mieux dotées en matériel et ressources humaines à pouvoir y répondre dans les délais impartis.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'illectronisme en France cause une véritable fracture et fragilise notre société ; c'est un constat indéniable. Dans un monde toujours plus connecté, avec une administration toujours plus numérisée qui laisse en marge trois Français sur cinq, avec des confinements successifs, qui ont accéléré le développement du télétravail, de l'école numérique à la maison ou encore de la télémédecine, la réduction de cette fracture doit devenir une de nos priorités nationales. Il y a quelques mois, la mission d'information du Sénat sur la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique, à laquelle j'ai participé, a permis de faire un état des lieux de la situation actuelle. du groupe RDSE, que nous examinons aujourd'hui, reprend une partie des 45 propositions alors formulées. Bien qu'elle ne règle pas tous les problèmes et présente quelques faiblesses juridiques identifiées par notre rapporteur, elle constitue une première pierre qui est à l'honneur du Sénat. Je partage avec mon groupe les préoccupations de son auteur visant à renforcer les instruments de lutte contre l'illectronisme et à faciliter l'accès aux services publics dématérialisés dans les territoires.

parmi les plus touchées par l'illectronisme. À ce sujet, je salue les amendements de notre collègue Philippe Mouiller, qui viennent compléter ce point. Des mesures qui me paraissent indispensables pour favoriser l'inclusion numérique des travailleurs sociaux, des élèves et des enseignants sont également proposées. instituée par la délégation aux entreprises sur les nouveaux modes de travail et de management, je ne peux que me féliciter de l'article 14 instaurant un crédit d'impôt au bénéfice des petites et moyennes entreprises, afin de favoriser la formation aux outils numériques des dirigeants et de leurs salariés. Nous savons que l'inégalité est grande devant le télétravail, mais aussi que la transformation numérique des entreprises est l'un des enjeux de la relance de leurs activités. Lutter contre l'illectronisme, ce sont de nombreux paramètres à faire avancer ensemble, car ils ne vont pas les uns sans les autres : haut débit, aide financière à l'accès au numérique et au matériel, meilleure ergonomie des sites et droit à l'erreur ne sont rien, si l'utilisateur n'en a pas la connaissance ou la maîtrise.